La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les explications de vote des groupes sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

était importante, parce qu'en matière pénale, nous avions également relevé la nécessité absolue d'une corrélation essentielle entre le prononcé de la peine et son exécution. Elle

Nous avons également conservé la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux, limité les procédures sans audience ainsi que la dématérialisation des procédures, sans négliger l'accès au juge pour tous les justiciables.

également prévu la présence de l'avocat lors des perquisitions, notamment en cas de flagrance. Très bien ! Nous avons maintenu le droit, pour le justiciable, de refuser le recours à la visioconférence, nous avons préservé la collégialité des travaux devant la chambre de l'instruction et nous avons supprimé

la création d'une peine générale d'interdiction du territoire français ; le relevé automatique de l'état de récidive ; la révocation automatique du sursis par une décision motivée de la juridiction ; enfin, le maintien des peines d'emprisonnement inférieures à un mois, afin d'éviter les effets de seuil. Cela montre à quel point le Sénat est attaché à la fermeté et à la clarté de la

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les corapporteurs, mes chers collègues, le groupe La République En Marche était, pour sa part, d'accord avec les objectifs que le Gouvernement avait exprimés en présentant ces projets de loi faire de la justice une priorité et mettre en oeuvre un vaste mouvement de réorganisation et de numérisation de celle-ci, en la dotant de moyens importants. Au cours de l'examen de ces textes, il est vrai que des dissensions sont apparues entre nous, notamment sur le divorce ou sur l'échelle des peines.

pour chacune des parties, de demander des mesures provisoires. Cette audience pouvait s'apparenter à l'audience de tentative de conciliation.

les textes qui nous réunissent de nouveau aujourd'hui ont donné lieu à beaucoup de points d'accord sur des mesures essentielles. Je pense à la mise en place d'un mode de saisine unique en matière civile, et des tribunaux de grande instance, ou encore à l'expérimentation du tribunal criminel départemental. Je pense également à la réforme des ordonnances d'injonction de payer, qui vise à centraliser le traitement

Sur ce dernier point, il est clair que les discussions doivent être encore plus poussées. L'aide juridictionnelle mérite une réforme d'ensemble nous faut examiner tous les paramètres de cette institution très importante pour notre justice, et non pas procéder, comme cela a été tenté à l'occasion de ces projets de loi, à des retouches partielles. L'aide juridictionnelle L'aide juridictionnelle mérite qu'on y consacre du temps et un projet global de réforme. Sur le parquet national antiterroriste, je regrette, au vu de l'importance du sujet, qu'aucun accord n'ait été trouvé. dit, le groupe La République En Marche ne s'opposera pas à ce que le débat se poursuive sur ces sujets à l'Assemblée nationale, dans le respect du bicamérisme. C'est la raison pour laquelle, malgré les divergences dont j'ai fait état, nous voterons en faveur de ces textes ainsi modifiés.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, messieurs les corapporteurs, mes chers collègues, il y a un an, presque jour pour jour, nous débattions ici du projet de redressement de la justice de la droite sénatoriale, conduite par Philippe Bas.

De manière générale, le projet du Gouvernement nous déçoit tant sur la forme que sur le fond. Une myriade d'articles protéiformes expriment un objectif dangereux : il s'agirait de redresser la justice en traitant l'embolie diagnostiquée de nos juridictions à coups de mesures gestionnaires et comptables. toujours la même logique, après la réforme du transport ferroviaire et avant celle des hôpitaux. Bien que vous vous en défendiez, madame la garde des sceaux- de bonne foi, je pense -, je peux vous assurer que la main invisible de Bercy n'épargne pas votre ministère, aussi régalien soit-il Sur la forme des débats, certes, nous nous réjouissons que la première lecture de ce texte ait fait honneur au Sénat. Nous nous interrogeons cependant sur la qualité de nos échanges, qui ont été

si nous nous félicitons de la majoration de 10 % de l'augmentation des crédits prévus pour la période 2018-2022, qui rétablit la trajectoire budgétaire adoptée par le Sénat l'année dernière, la question de la ventilation de ces moyens continue à susciter des Nous constatons ainsi que l'augmentation des crédits proposée s'inscrit dans la même orientation que celle de ces dernières années : l'impact de cette progression, telle que cela est suggéré, est largement réduit pour les services judiciaires ou l'accès à la justice, puisque le programme de l'administration pénitentiaire l'absorbe en grande partie. Sur la procédure Sur la procédure civile, nous nous réjouissons des modifications apportées par notre commission des lois ; son travail d'amélioration dans l'objectif de « mieux protéger les personnes vulnérables Nous saluons le travail de nos corapporteurs dans ce sens, ainsi que leur intention de combattre la déjudiciarisation dont était pétri le texte du Gouvernement dans un seul et simple souci économique. Nous espérons que leurs modifications résisteront aux lectures à venir. Nous nous félicitons notamment de la conservation par la commission des lois de la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux, que le texte gouvernemental supprimait. Nous approuvons aussi la suppression de la dématérialisation de certaines procédures lorsqu'elle se faisait au détriment de l'accès au juge pour les justiciables. Sur la procédure pénale, quelques apports des corapporteurs ne sont pas négligeables non plus. Nous partageons leur constat d'un renforcement excessif du pouvoir du parquet. De ce fait, nous saluons la conservation de l'obligation de présentation au procureur pour la prolongation de garde à vue et celle de l'accord de la personne mise en cause pour la visioconférence lorsque le juge statue sur la détention provisoire. Saluons aussi la limitation de l'extension à de nouvelles infractions des techniques d'enquête intrusives pour la vie privée, et surtout le maintien de la collégialité des travaux de la chambre de l'instruction. Nous regrettons néanmoins l'adoption d'un certain nombre d'autres mesures qui justifient notre opposition. Par exemple, l'expérimentation du tribunal criminel départemental porte atteinte selon nous à un fondement de notre justice républicaine, les jurés populaires l'extension de l'amende forfaitaire délictuelle ne fait quant à elle que poursuivre l'échec de la politique répressive en matière de lutte contre la drogue, politique à l'oeuvre depuis trop longtemps et particulièrement délétère, notamment pour nos mineurs. Sur l'efficacité et le sens des peines en matière de justice pénale, messieurs les corapporteurs, vos propositions nous inquiètent et témoignent de l'urgence qu'il y a à réfléchir sérieusement sur le sens de la peine et l'échelle des peines. Je vous rappelle, mes chers collègues, que la peine a trois vocations : punir, protéger la société, et réinsérer. Dans ce texte, la réinsertion n'a que très peu de place ; au contraire, la peine n'est envisagée presque que sous l'angle de la punition. En outre, l'unique peine considérée comme possible est la prison, comme s'il n'existait que celle-ci. Sur l'organisation des juridictions, enfin, point crucial d'accord entre le Gouvernement et la droite sénatoriale, quel que soit le nom qui sera finalement retenu pour les tribunaux uniques de première instance, leur création poursuit la logique qui consiste à englober les tribunaux d'instance dans les tribunaux de grande instance. Cela est pour nous révélateur de la déshumanisation de la justice, que l'on engage, notamment, en s'attaquant à sa proximité avec le justiciable. La suppression à venir des tribunaux d'instance, en en commençant par leur dévitalisation, n'ira que dans ce sens. Nous le regrettons amèrement. En effet, la justice, je le répète, fait l'objet d'une politique publique bien particulière, car elle est essentielle à notre État de droit : sans son bon fonctionnement, c'est toute la société qui s'effondre Sur les ajouts de la commission des lois, et notamment sur le point de l'accès à la justice, faire précéder toute demande d'aide juridictionnelle de la consultation d'un avocat ajoute selon nous un obstacle supplémentaire au parcours du justiciable qui souhaite saisir la justice et qui n'en a pas les moyens. De plus, confier aux avocats, qui sont des acteurs privés, une mission qui relève de l'autorité de l'administration, et ce dans le seul objectif de réaliser des économies, est pour nous inadmissible. S'attaquer à l'aide juridictionnelle, c'est s'attaquer à la fonction essentielle de la justice, à savoir rétablir l'égalité des armes entre les parties. L'aide juridictionnelle est un moyen précieux d'accéder à la même justice pour tous. Pour toutes ces raisons, et également parce que le Sénat, malgré sa fidélité à son rôle de défenseur des libertés individuelles, n'a modifié le texte qu'à la marge sans rien changer à son économie générale, nous voterons contre ces deux projets de loi.

la justice est le parent pauvre, l'institution à laquelle nous n'avons pas, dans le passé, donné suffisamment de moyens ; chaque gouvernement s'en préoccupe de manière plus ou moins heureuse.

C'était la réforme de la carte judiciaire, qui laisse encore des doutes dans les esprits ; madame la garde des sceaux, vous le savez bien. C'était aussi la loi

Sous le précédent quinquennat, la garde des sceaux, Mme Taubira, avait lancé les états généraux de la justice. Ce grand débat aurait pu inspirer le gouvernement actuel,

faire des économies, au risque d'entraîner une déjudiciarisation et une déshumanisation. Or nos concitoyens ont besoin de la justice. Je reprends l'exemple du divorce. Certes, lorsque les époux sont d'accord, ils n'ont pas besoin d'aller voir le juge

en lieu et place de la contrainte pénale, non pas la détention à domicile, qui était un moyen d'organiser l'emprisonnement, mais la probation ; cette dernière est une synthèse entre le sursis avec mise à l'épreuve, qui ne fonctionne pas,

je commencerai par un satisfecit, pour saluer le climat apaisé et constructif dans lequel ces deux textes ont été examinés. Compte tenu de l'importance des sujets abordés et de la mise en oeuvre de la procédure accélérée,

Nos débats ont souvent permis de souligner, en matière pénale notamment, qu'il existe une volonté commune de changer de modèle. Les hésitations qui demeurent portent essentiellement sur l'anticipation des effets directs et indirects des dispositifs que nous élaborons. Je pense notamment à la révision de l'échelle des peines correctionnelles, à la peine autonome de probation, ou encore à l'expérimentation d'un tribunal criminel. La justice que nous défendons, au groupe du RDSE, est une justice accessible, lisible et impartiale, dont l'impartialité est garantie soit par le statut de fonctionnaire du magistrat rendant justice, soit par la reconnaissance par ses pairs. À ce stade, ces deux textes contiennent donc des éléments de nature à nous réjouir, mais également des dispositions ambiguës ou plus contestables. Les nouvelles technologies de communication sont certes devenues des outils incontournables pour une majorité de Français. elles peuvent produire des effets ambivalents en matière de justice. Elles permettent sans doute d'accélérer la résolution de conflits pour une partie de la population. Toutefois, dans le même temps, elles réduisent l'accès à la justice de nos concitoyens victimes de la fracture numérique. C'est pourquoi nous restons très dubitatifs quant à l'extension à court terme de la dématérialisation des procédures. Il en va de même des modes alternatifs de règlement des différends, qui sont des outils de pacification sociale intéressants, à condition qu'ils ne soient pas systématiquement rendus obligatoires ni uniquement utilisés afin de réguler le stock de contentieux.

Ce constat semble illustrer l'existence d'un stock constant de litiges pour lesquels l'intervention du juge sera toujours nécessaire, en raison de la confiance que le justiciable place dans l'autorité judiciaire. Nous craignons plus encore que les nouvelles dispositions introduites en commission des lois, au sujet de l'aide juridictionnelle, ne menacent l'accès au juge. Nous pensons, en particulier, à nos concitoyens les plus vulnérables, ceux qui ne peuvent s'acquitter d'un droit de timbre ou qui renoncent à recourir à un avocat avant l'obtention de l'aide juridictionnelle. De plus, nous regrettons qu'un certain nombre de propositions que nous avions formulées n'aient pas été inscrites dans ces je songe à la revalorisation du statut de juriste assistant. Je l'évoquais lors de la discussion générale : partout où elle recule, la collégialité de la décision de justice doit être compensée par une collégialité de cabinet, qui sorte le juge de sa solitude de juge unique. Les assistants et greffiers qui assistent les magistrats ne doivent pas être perçus comme de simples délégataires des tâches les plus ennuyeuses. Leurs fonctions doivent s'inscrire dans une trajectoire professionnelle de long terme au sein des juridictions. au sujet de la prise en charge juridique des mineurs isolés étrangers, nous avons entendu vos réponses. Mais nous considérons que l'urgence de leur situation justifie d'apporter des solutions dès à présent. Beaucoup d'entre eux sont des adolescents aujourd'hui. Il n'est pas concevable de reporter le règlement de leur situation dans un ou deux ans. Nous exprimons les mêmes regrets quant au rejet des amendements de notre collègue Françoise Laborde, visant à assurer une meilleure prise en compte des victimes de violences conjugales.

d'insécurité., alors que la réforme de la carte judiciaire a suscité beaucoup d'inquiétudes dans les territoires, les solutions proposées par nos corapporteurs sont rassurantes, à commencer par l'abandon de la spécialisation des chambres détachées et des cours d'appel. Néanmoins, comme l'a souligné notre collègue Sophie Joissains, une chambre détachée restera toujours plus facile à fermer qu'une juridiction. Nous resterons donc particulièrement vigilants sur ces points, car nous nous opposerons toujours aux effets indésirables de la métropolisation, qui consisteraient à faire des métropoles la seule référence des cartes administratives au détriment de l'échelle départementale, laquelle est beaucoup plus humaine. La réussite de la réforme de la justice dépendra aussi de la confiance des agents envers les outils que nous mettons à leur disposition. C'est pourquoi il est si difficile de réformer des institutions qui fonctionnent bien, comme les tribunaux d'instance ou les cours d'assises. Vous vous y êtes pourtant attelée, madame la garde des sceaux, et il faut saluer l'approche globale que vous avez voulu suivre pour votre réforme. D'autres outils judiciaires sont en plus mauvais état en avons conscience, il est urgent de rénover le parc carcéral, et avec lui, le sens de la peine. Grâce au travail accompli par la Chancellerie et par la commission des lois, le débat a permis de faire émerger un consensus autour de la nécessité de marginaliser l'emprisonnement en matière délictuelle. Il importe que la prison ne soit plus perçue comme un « rite de passage », par lequel les jeunes délinquants vont s'endurcir dans des conditions matérielles indignes, aux côtés de condamnés plus aguerris et parfois radicalisés. Il importe également de sortir de prison les personnes dont la santé exige des soins psychiatriques lourds. C'était l'objet des amendements que nous avions déposés avec notre collègue Nathalie Delattre. Certaines propositions, comme l'atténuation du principe de séparation des prévenus et des condamnés en vue d'optimiser l'occupation dans les maisons d'arrêt, nous semblent particulièrement pertinentes. Le sens doit enfin guider notre plume quand nous légiférons sur les travaux d'intérêt général menés à des fins de réadaptation : nous avons bon espoir que l'agence créée par le texte permette le développement de cette sanction, à condition qu'elle soit effectivement mise au service de la collectivité.

Monsieur le président, madame le ministre, chers collègues, ces textes présentent des aspects positifs, mais aussi des aspects beaucoup plus discutables. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai.

honnête et cohérente. Et ce qui est fait pour les cours d'appel vaut aussi pour d'autres tribunaux.

Monsieur le président, Monsieur le président, madame la garde des sceaux, messieurs les corapporteurs, mes chers collègues, l'ambition des deux textes qui vont être mis aux voix dans un instant est-elle à la hauteur de leur intitulé ? Est-ce une « réforme pour la justice » ? Est-ce bien l'électrochoc dont notre système a besoin ? À nos yeux, avant que le Sénat ne s'en saisisse, la réponse était négative. Nous avions un florilège de mesures, souvent intéressantes d'ailleurs, mais non une réforme ambitieuse. Nous avions un catalogue assez fourni que l'on aurait pu appeler « diverses dispositions en matière de justice ». Vous avez pu le constater, madame la garde des sceaux, le Sénat n'a pas été avare de propositions lors des semaines d'examen des deux projets de loi, et pour cause : notre commission des lois est mobilisée sur ce sujet depuis des années, notamment pour ce qui concerne son aspect budgétaire, qui ne règle pas tout, évidemment, mais qui est fondamental. Notre collègue Yves Détraigne, dont je salue l'implication dans ce dossier, nous alerte inlassablement lors de chaque projet de loi de finances sur de nombreux problèmes : le manque criant de moyens, l'état de délabrement des juridictions, l'insalubrité de nombreuses prisons, ou encore les moyens informatiques d'un autre âge avec lesquels greffiers et magistrats Nous avons donc modifié l'article 1 du projet de loi, qui fixe la programmation pluriannuelle, conformément à ce que nous estimons indispensable au redressement de notre justice. La réflexion du Sénat sur le sujet ne se limite pas à cet aspect financier qui, je le répète, ne règle pas tout. Nos corapporteurs se sont appuyés sur les travaux de la mission d'information sénatoriale sur le redressement de la justice, lancée en 2016. Celle-ci avait abouti à pas moins de 127 propositions, et elle a conduit à l'adoption par le Sénat de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice, le 24 octobre 2017.

claire : tenter de rétablir, point par point, presque obstinément, le texte initial. Je reconnais que vous avez toujours cherché à argumenter vos positions, et que la qualité de nos débats mérite d'être saluée. Oui ! Mais, au total, qu'en est-il du travail parlementaire ?

quelques mots. L'une des orientations du projet de loi, qui ne fait d'ailleurs qu'accentuer un phénomène semblant inéluctable depuis plusieurs années, c'est l'augmentation des pouvoirs des magistrats du parquet. Nous n'y sommes pas opposés par principe, mais il faut être prudent à ce sujet. On ne peut occulter le fait que les parquetiers ne constituent pas une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La France a déjà subi plusieurs condamnations à ce titre. Or cette situation ne pourra pas s'améliorer tant que nous n'aurons pas apporté des garanties supplémentaires d'indépendance statutaire en révisant notre Constitution ... Exactement ! C'est une Notre commission a fait, sur ce volet du texte, un important travail, fidèle à la tradition de défense des libertés individuelles à laquelle la Haute Assemblée est attachée. Les modifications votées sur l'initiative de nos collègues Buffet et Détraigne ont permis de préserver un équilibre entre l'efficacité dans la recherche des auteurs d'infractions, les libertés et les droits de la défense. Les travaux en séance ont permis d'ajouter au projet de loi ordinaire de nombreuses autres dispositions que nous avions adoptées en 2017, comme la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les étrangers coupables de délits et crimes punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ou encore la suppression du principe de l'attribution automatique de crédits de réduction de peines aux condamnés détenus. Nous nous félicitons de ces modifications et espérons qu'elles seront adoptées par l'Assemblée nationale.

élus de notre groupe veilleront à ce que cette réforme ne conduise, ni aujourd'hui ni demain, à la fermeture d'implantations judiciaires. Mes collègues et moi-même sommes en effet extrêmement attachés au maintien de tous ces lieux de justice, au nom de l'exigence de proximité pour le justiciable. vous l'aurez compris, une majorité de notre groupe est convaincue que le travail du Sénat a permis de redonner à cette réforme le souffle et la vision qui lui faisaient défaut. Cette transformation a été rendue possible par le travail de nos deux corapporteurs, François-Noël Buffet et Yves Détraigne,

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, messieurs les corapporteurs, mes chers collègues, aujourd'hui procéder au vote, d'une part, du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, de l'autre, du projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions. Ces textes visent, selon le Gouvernement, à « rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice ». Ils ont également pour Je souhaite à nouveau mettre l'accent sur la situation de notre justice, qui ne s'améliore pas, et pour cause : le problème de fond est évidemment celui des moyens. Oui, la justice de notre pays est dans un état critique aujourd'hui, car elle souffre d'un manque d'investissement prolongé. Des délais de jugement qui s'allongent, une situation chronique de sous-effectif liée aux vacances de postes, un système illisible d'exécution des peines, en vertu duquel la peine exécutée n'est, souvent, pas la peine prononcée, une surpopulation carcérale chronique

Je souhaite également relever à cette tribune la qualité des travaux menés par nos collègues François-Noël Buffet et Yves Détraigne. Sur leur initiative, la commission a inséré dans ces projets de loi plusieurs dispositions issues de la proposition de loi d'orientation et de programmation et de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice, déposées au Sénat par Philippe Bas, président de la commission des lois, à l'issue des travaux de la mission d'information sur le redressement de la justice. Les textes qui sont soumis au vote aujourd'hui couvrent un champ très vaste. Ils balayent notamment le droit civil, le droit pénal, la procédure pénale et l'organisation judiciaire, les nombreuses modifications introduites par les deux corapporteurs ont permis de les améliorer. Ainsi, en matière budgétaire, la commission a demandé un effort plus important, à la hauteur des enjeux du redressement de la justice. En matière de justice civile, elle a amélioré l'efficacité et la rapidité des procédures tout en veillant à la protection des personnes vulnérables par la suppression ou l'encadrement de certaines mesures.

En matière d'organisation judiciaire, elle a clarifié la réforme, avec la création du tribunal de première instance, tout en veillant au maillage territorial et à la proximité de l'institution judiciaire. Je me réjouis également que la commission ait restauré la crédibilité du prononcé et de l'exécution des peines en supprimant tout examen obligatoire des peines d'emprisonnement aux fins d'aménagement, et qu'elle ait fait de la probation une peine autonome, que le juge peut prononcer, le cas échéant, en complément d'une peine d'emprisonnement. Je me félicite enfin que la commission ait supprimé le caractère automatique de la libération sous contrainte aux deux tiers de la peine. Les débats en séance ont permis de nombreux apports intéressants. Parmi ceux-ci, je tiens à citer la possibilité donnée aux victimes d'agression d'être informées du statut carcéral de leur agresseur et des conditions de sa sortie d'incarcération ; la création d'une peine complémentaire générale d'interdiction du territoire français pour les étrangers coupables de délits et crimes punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement la suppression du principe de l'attribution automatique de crédits de réduction de peines aux condamnés détenus ; l'expérimentation d'un vote par correspondance pour les personnes détenues ; l'organisation d'un « isolement électronique » des détenus dans leur cellule la possibilité de procéder en prison, sur les visiteurs, à toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l'établissement. Madame la ministre, mes chers collègues, l'état dans lequel se trouve la justice de notre pays nécessite des mesures fortes, urgentes et efficaces. Ces deux textes modifiés par le Sénat apportent de réelles réponses

il va être procédé, dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement, au scrutin public solennel sur l'ensemble du projet de loi

La séance est suspendue.

Le scrutin est ouvert.

pour remercier le Sénat de la qualité des débats qui se sont tenus durant ces deux dernières semaines. J'adresse ces remerciements tout d'abord au président de la commission des lois, M. Philippe Bas ainsi qu'aux deux corapporteurs, MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne,

Ces groupes font preuve d'une violence aveugle, mais ils ont une cible : nos forces de l'ordre, nos institutions, en somme, la République ! Ces Black Blocs, comme on les appelle, ne s'en prennent pas seulement aux biens, mais d'abord aux personnes dépositaires de l'autorité publique, à coup de fusées, de barres de fer, de battes de base-ball et d'armes en tout genre. Lorsqu'ils cherchent à blesser, voire pire, nos policiers ou nos gendarmes,

; elle doit casser leur logique de haine, en particulier de haine anti-flics, qui est inacceptable et insupportable. Notre rôle de législateur est d'opposer à cette loi du plus fort la force de la loi. Or, aujourd'hui, la loi présente trop de

L'objectif de cette proposition de loi est donc de renforcer notre législation afin de l'adapter aux modes d'action de ces groupes. À cette fin, je vous propose que la loi confère aux responsables de la sécurité publique

du volet répressif, je propose de punir sévèrement d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende le fait de dissimuler son visage pendant une manifestation et de cinq ans de prison et de 4 500 euros d'amende le fait de porter une arme lors d'une manifestation sur la voie publique. Mes chers collègues, à qui fera-t-on croire que cacher son visage dans ces manifestations hyperviolentes n'est qu'une manière de se protéger contre les coups de soleil ? de soleil ? Enfin, les dégâts matériels causés par ces individus sont parfois considérables et c'est le contribuable qui paye. Il faut mettre fin à ce régime d'irresponsabilité et permettre enfin à l'État de faire payer à ces délinquants le coût de leurs violences. Le principe doit être simple et efficace : celui qui casse paye. casse paye. Mes chers collègues, nous sommes tous attachés au droit de manifester. Il s'agit d'une liberté absolument fondamentale que nous devons renforcer.

au désordre créé par ces violences ; notre devoir est de refuser que la République soit asservie par ceux qui se servent des manifestations pour casser, pour agresser, pour créer le chaos dans nos rues. Nous ne devons Nous ne devons pas rester désarmés, mes chers collègues, il faut agir, nous en avons les moyens ! La parole est

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, depuis quelques années, un grand nombre de manifestations sur la voie publique sont émaillées de violences et de dégradations d'une particulière gravité, qui nuisent au libre exercice du droit de manifester. Ces violences et ces dégradations sont le fait de groupuscules ultra-violents, notamment désignés sous le terme de Black Blocs, qui se créent et disparaissent à l'occasion de chaque manifestation. Ils ont en effet pour unique objectif de se fondre dans les cortèges pacifiques pour commettre des dégradations et des violences. Ainsi, 1 200 Black Blocs se sont infiltrés dans les cortèges de la manifestation du 1 mai dernier à Paris et ont provoqué, par des actes d'une violence inouïe, des dégâts et dégradations d'une ampleur considérable. Je puis en témoigner, car je me trouvais alors en face de l'hôpital Necker-Enfants malades qui a été vandalisé. Il serait erroné de dire que nous sommes complètement démunis face à ces phénomènes de violence. Au cours des vingt dernières années, le législateur a en effet renforcé le cadre juridique du maintien de l'ordre en créant de nouveaux outils destinés à prévenir le plus en amont possible les débordements dans les manifestations publiques. L'autorité administrative a été ainsi dotée de nouvelles prérogatives, parmi lesquelles la possibilité, lors des manifestations, de recourir à la vidéoprotection ou d'interdire le port et le transport d'objets pouvant constituer une arme le législateur a, de plus, renforcé l'arsenal répressif, en créant une série d'incriminations spécifiques destinées à sanctionner les faits troublant ou susceptibles de troubler l'ordre public commis à l'occasion d'une manifestation, notamment

La judiciarisation du maintien de l'ordre et la sanction des actes délictuels commis à l'occasion des manifestations se heurtent en effet, dans la pratique, à des difficultés opérationnelles majeures. Les contraintes liées au maintien de l'ordre nuisent très souvent à la qualité des procédures diligentées ou à la collecte des preuves qui permettraient d'imputer les infractions constatées aux personnes interpellées. De plus, la présentation en masse de personnes interpellées aux autorités de police judiciaire n'est généralement pas compatible avec le cadre juridique inhérent au placement en garde à vue. Or, faute d'éléments de preuve ou de procédures solides, les parquets sont trop souvent contraints de prononcer des classements sans suite. Les difficultés à engager des procédures judiciaires sont exacerbées lorsqu'il s'agit de Black Blocs, car ceux-ci recourent à des modes d'action spécifiques, conçus pour entraver l'intervention des pouvoirs publics. Il est ainsi particulièrement difficile d'interpeller les Black Blocs au cours d'une manifestation, en raison de leur capacité à se mêler rapidement aux manifestants pacifiques, après avoir abandonné, voire brûlé, leurs équipements. Il n'est pas plus aisé de les identifier, au moyendes images de vidéoprotection, car ils agissent masqués et vêtus de noir. Sans avoir pour ambition de résoudre l'ensemble des difficultés soulevées, qui relèvent pour partie de l'organisationnel, la proposition de loi sur laquelle nous sommes appelés à nous prononcer aujourd'hui tend à apporter une première série de réponses. Elle prévoit des mesures fortes, destinées à faciliter l'action des pouvoirs publics à l'égard de ces groupuscules ultra-violents. Elle s'inscrit dans un mouvement déjà engagé par le législateur au cours des dernières années, qui privilégie une logique chirurgicale, afin d'écarter de la foule les individus perturbateurs ou les casseurs, tout en permettant aux cortèges pacifiques de continuer à manifester. Je regrette d'ailleurs, monsieur le secrétaire que la commission des lois n'ait pas été en mesure de recevoir l'avis de la préfecture de police de Paris- pourtant essentiel en ce qui concerne le maintien de l'ordre -, car les réponses écrites que nous attendions n'avaient pu être validées au plus haut niveau, faute de ministre La proposition de loi comporte trois volets, que la commission des lois a approuvés et sécurisés, afin de prévenir efficacement les atteintes à l'ordre public, dans le respect des droits et des libertés constitutionnellement garantis. Son premier volet est préventif. Il vise à doter l'autorité administrative de nouveaux instruments destinés à prévenir, le plus en amont possible, l'infiltration des manifestations pacifiques par des individus violents. En premier lieu, il confère au préfet la possibilité de diligenter, par arrêté, un contrôle des effets personnels des passants dans le périmètre ou aux abords immédiats d'une manifestation, lorsqu'il existe des risques de troubles graves à l'ordre public. Ces contrôles comprendraient des palpations de sécurité et des fouilles de sacs et ne pourraient s'effectuer qu'avec le consentement des personnes contrôlées. Il n'est en revanche pas prévu que des contrôles d'identité et des fouilles de véhicules puissent être réalisés. Il s'agit, à quelques différences près, d'une extension des périmètres de protection que nous avions créés dans la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. En deuxième En deuxième lieu, la proposition de loi vise à autoriser les préfets à prononcer, à l'encontre de toute personne susceptible de représenter une menace d'une particulière particulière gravité pour l'ordre public, une interdiction de participer à une manifestation, assortie, le cas échéant, d'une obligation de pointage auprès d'un représentant de l'autorité publique. L'interdiction de manifester n'est pas inconnue dans notre droit, mais elle n'existe, actuellement, qu'à titre de peine complémentaire, pour une durée de trois ans. Il s'agirait, ici,

dans son rapport rédigé au nom de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative au maintien de l'ordre. Enfin, de manière conséquente, la proposition de loi prévoit la création d'un fichier national recensant l'ensemble des mesures d'interdiction de manifester, qu'elles soient prononcées dans un cadre judiciaire administratif, afin d'en faciliter le suivi, notamment à l'occasion des contrôles de police. Ces mesures confèrent à l'autorité préfectorale de larges prérogatives, mais elles ont le mérite de permettre d'écarter, dès avant la manifestation, les individus animés par la seule volonté de commettre des dégradations. Il ne s'agit en aucun cas de porter atteinte à la liberté de manifester, mais au contraire d'en garantir le libre exercice par les manifestants pacifiques, en évitant qu'ils ne soient pris en otage par une poignée d'individus désireux de se livrer à une action violente. L'adaptation de ces mesures présenterait également l'avantage de compléter l'arsenal juridique à la disposition de l'autorité préfectorale et, ainsi, de permettre une réponse graduée en cas de menaces à l'ordre public. Il est préférable, j'en suis convaincue, d'empêcher quelques individus de manifester plutôt que d'interdire la tenue d'une manifestation. Dans cette perspective, la commission a complété

Le deuxième volet de la proposition de loi est répressif et vise à sanctionner plus sévèrement les auteurs de violences et de dégradations dans les manifestations. Il comprend plusieurs dispositions pénales, auxquelles la commission des lois a apporté quelques modifications pour en assurer l'intelligibilité et la clarté.

puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Ensuite, la proposition de loi élargit l'infraction de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme, afin de viser le port non seulement d'une arme, mais aussi d'une arme par destination, de fusées et d'artifices. Enfin, plusieurs dispositions renforcent et élargissent la peine complémentaire d'interdiction de manifester. Le troisième volet de la proposition de loi consiste en une réforme, prévue à l'article 7, du régime de la responsabilité civile applicable en cas de dommages causés dans le cadre d'une manifestation. a été entièrement réécrit par la commission des lois, qui a souhaité répondre à l'objectif visé par les auteurs de la proposition de loi- mieux responsabiliser les auteurs de dégâts -, tout en garantissant un régime juridique viable et applicable sur le plan opérationnel. Le dispositif initial instaurait une présomption de responsabilité civile collective des personnes condamnées pénalement pour des infractions commises à l'occasion d'une manifestation, y compris pour des dommages sans lien avec la faute commise par chacune de ces personnes. Cette disposition appelait, tout d'abord, d'importantes réserves constitutionnelles, dans la mesure où elle aurait permis de reconnaître la responsabilité d'un individu pour des dommages qu'il n'a pas causés. Elle risquait ensuite d'affaiblir la protection des victimes. En effet, le régime actuel de responsabilité sans faute de l'État pour tous les dommages commis lors des manifestations garantit le remboursement des victimes.

En précisant et complétant les dispositions de cette proposition de loi, la commission des lois a abouti, je crois, à un équilibre satisfaisant entre les exigences de sécurité publique et la nécessaire protection des droits et libertés.

monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur,

des symboles de la République, du mobilier urbain ou des magasins ou enseignes qui seraient les symboles d'une société moderne. Pour les prévenir, pour garantir l'exercice de la liberté de manifester en permettant à chaque citoyen, s'il le souhaite, de se rendre sans crainte sur les lieux d'une manifestation, les préfets font appel aux membres des compagnies républicaines de sécurité et aux militaires de la gendarmerie mobile, ainsi qu'à l'ensemble des effectifs de sécurité publique, de gendarmerie départementale et, pour les nombreuses manifestations qui se déroulent dans la capitale, de la préfecture de police de Paris.

aux opérations d'évacuation menées au sein de plusieurs facultés à Paris et dans certaines grandes agglomérations, aux nombreuses journées nationales de mobilisation et, bien sûr, aux manifestations du mois de mai évoquées il y a quelques instants et à ces images choquantes de Black Blocs encagoulés en tête de la manifestation. en tête de la manifestation. Toujours en première ligne, particulièrement exposées, nos forces de sécurité risquent leur intégrité physique dans ces opérations compliquées, où certains cherchent constamment à les pousser à la faute, sous le regard permanent des médias et des réseaux sociaux. Comme vous le savez, mon expérience passée m'a conduit à diriger de nombreux services d'ordre public : je suis donc bien placé pour en témoigner. Le ministre de l'intérieur en est également parfaitement conscient.

Il avait alors présenté plusieurs axes de travail, que nous sommes en train de décliner sur le terrain de manière opérationnelle, pour mieux prévoir, mieux préparer, mieux anticiper et mieux contrôler ces manoeuvres d'ordre public-

Il est en effet de notre responsabilité de mieux anticiper les trois temps d'une manifestation- l'avant, le pendant et l'après -, pour mettre un terme au sentiment d'impuissance que certains ont pu ressentir lorsque les pouvoirs publics n'ont pas été en mesure de faire cesser les agissements de personnes venues spécialement pour en découdre, commettre des violences et casser. L'absence de dispositif administratif spécifique d'interdiction individuelle de manifester et l'absence de poursuites pénales ou de condamnation des fauteurs de troubles suscitent légitimement une forme d'incompréhension chez nos concitoyens. C'est pourquoi un groupe de travail spécifique, composé de juristes et d'opérationnels, a été installé par le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice, pour convenir des moyens les plus simples et les plus efficaces de mieux détecter, interpeller, puis sanctionner les fauteurs de troubles.

Il en est ainsi de la création d'un périmètre de protection permettant le contrôle des personnes pendant les six heures précédant une manifestation, de la possibilité pour l'autorité administrative d'interdire à toute personne susceptible de se livrer à des violences de participer à une manifestation à une manifestation et de la création d'un fichier des interdictions de manifester. Je pense également à la transformation de la contravention de la cinquième classe de dissimulation illicite du visage à l'occasion d'une manifestation en un délit, permettant une signalisation de la personne, un placement en garde à vue et l'engagement d'une procédure rapide,

D'autres dispositifs, en revanche, n'atteignent pas, à mes yeux, l'objectif assigné à cette proposition de loi. C'est notamment le cas des articles 5 et 6 du texte. L'article 5 procède à une simple réécriture du délit de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme. Cette modification ne nous semble pas nécessaire, dans la mesure où le port ou l'introduction d'armes par destination lors d'une manifestation peut déjà être réprimé par l'infraction prévue à l'article 431-10 du code pénal, qui sanctionne le fait de participer à une manifestation en étant porteur d'une arme. Pour ces raisons, introduire des exemples d'armes dans la loi n'est pas souhaitable : cela risquerait d'entraîner un affaiblissement du droit et de soulever des difficultés d'interprétation de celui-ci. De même, l'article 6 ne pourra recueillir l'avis favorable du Gouvernement. Il vise à étendre des peines complémentaires d'interdiction de séjour, la privation des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction de détenir une arme pendant cinq ans et la confiscation de l'arme au nouveau délit de dissimulation du visage aux abords d'une manifestation, ainsi qu'au délit d'organisation d'une manifestation sans déclaration préalable. Or la possibilité de prononcer de telles peines pour ces délits faiblement réprimés semble disproportionnée au regard de la peine encourue.

Il ne s'agit pas pour le Gouvernement de rejeter en bloc cette proposition de loi, uniquement parce qu'elle serait défendue par l'opposition, mais d'avoir, pendant ces débats parlementaires, la possibilité d'un premier échange permettant de parvenir, dans quelques mois, à la rédaction d'un texte répondant au mieux aux attentes des praticiens : policiers, gendarmes, agents de police judiciaire et magistrats. cadre rénové, nos concitoyens puissent exercer la liberté essentielle qu'est le droit de manifester en toute sécurité, en sachant que l'ordre public est préservé et que les forces de sécurité intérieure disposent des outils juridiques nécessaires pour les protéger, se protéger et mettre à la disposition de la justice les fauteurs de troubles ! La parole

la proposition de loi soumise à notre examen a pour objectif de prévenir les violences lors des manifestations et de sanctionner leurs auteurs. Elle fait écho à celle de M. Courtial, déposée le 3 mai dernier, qui vise à interdire la dissimulation du visage lors d'une manifestation sur la voie publique. Nous sommes tous d'accord : les violences qui accompagnent régulièrement les manifestations discréditent le mouvement social et rendent inaudible le message porté par ceux qui y participent. Elles sont à condamner fermement et le professionnalisme dont font preuve les forces de l'ordre en pareil cas doit être salué.

On pourrait mentionner aussi les violences en marge des mouvements contre le contrat d'insertion professionnelle en 1994, le contrat première embauche en 2006- à l'époque, 187 personnes avaient été interpellées -et la loi Travail en 2016. Faire remonter cette violence aux manifestations du mois de mai ou, généreusement, à celles qui ont eu lieu sous le précédent quinquennat- mais personne ne s'aventurerait à faire cette confusion au sein de notre assemblée ... -serait donc parfaitement injuste. Parler de défaillance de l'actuel gouvernement le serait tout autant, convenons-en tous. Il serait donc inutile de chercher à politiser nos débats, d'autant que, fort heureusement, de nombreux rassemblements se déroulent encore dans le calme, comme en témoigne la Marche pour le climat de septembre dernier. La proposition de loi, dans sa rédaction initiale, présentait des risques importants pour les libertés individuelles. S'il est vrai que la commission des lois a cherché à sécuriser le texte afin de prévenir efficacement les atteintes à l'ordre public dans le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis, il me semble que l'équilibre n'a pas été tout à fait trouvé. La mesure qui consiste à donner la possibilité aux préfets d'interdire, par arrêté, à toute personne susceptible de représenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public de participer à une manifestation mérite d'être réétudiée.

Je pense à l'extension, aux abords immédiats d'une manifestation, de l'infraction de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme au fait d'introduire, de détenir ou de faire usage de tout objet susceptible d'en constituer une et, plus encore, à la sanction de la tentative même de ces délits, introduite par la commission des lois. Je pense également à l'extension du champ de la peine complémentaire d'interdiction de manifester.

Enfin, si, dans sa rédaction initiale, la proposition de loi instaurait une présomption de responsabilité civile collective en matière de dommages causés à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique, la commission des lois a fait le choix de maintenir le régime de responsabilité sans faute de l'État, tout en donnant à celui-ci la possibilité d'exercer une action récursoire contre les personnes condamnées pour les violences ou dégradations à l'origine des dommages. La question de l'effectivité de l'exercice de l'action récursoire reste posée, eu égard à l'état de solvabilité des personnes concernées. Au total, malgré le travail de qualité accompli par Mme la rapporteur, cette proposition de loi présente encore des risques élevés pour les libertés individuelles.

l'arsenal législatif déployé ces dernières années pour lutter contre la violence dans les manifestations est colossal. Mme Troendlé l'a rappelé en présentant son rapport : les prorogations successives de l'état d'urgence entre 2015 et 2017 les lois antiterroristes qui ont suivi ont largement contribué à alimenter cet arsenal. À tel point qu'Amnesty International a publié, le 31 mai 2017, un rapport intitulé.

question l'efficacité de ces mesures, pourtant nombreuses. C'est pourquoi ils proposent de les compléter. Au préalable, je rappelle, s'il en était besoin, que tous les membres de mon groupe condamnent l'action des Black Blocset de tout groupe troublant les manifestations pacifiques. Nous condamnons toutes les violences et dégradations dans l'espace public Ces individus portent atteinte d'abord aux manifestants eux-mêmes- nous savons de quoi nous parlons -et au droit de ceux-ci à manifester. Eh oui ! Leurs agissements nuisent surtout aux messages véhiculés et aux revendications légitimes des manifestants, bien souvent relégués au second plan par les médias, qui se focalisent généralement plus volontiers sur les débordements que sur le fond de la colère des manifestants. À cet égard, je m'interroge sur le fait qu'aucune des forces organisatrices de manifestations n'ait été auditionnée par Mme la rapporteur. Je les ai reçues ce matin, ma

Nous nous interrogeons en outre sur l'unique justification de cette proposition de loi visant clairement à restreindre le droit de manifester : la violence qui s'accroîtrait. Dans une interview donnée au à la suite des manifestations contre la loi Travail, Olivier Cahn, chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales, expliquait expliquait que le niveau de violence des manifestations en France avait baissé, malgré quelques débordements individuels. « Le niveau de violence a même eu tendance à baisser depuis les années 1970-1980 », constatait-il, en faisant parallèlement observer que, « structurellement, le maintien de l'ordre s'est durci ces dernières années en France, alors qu'à l'étranger la tendance est à la désescalade ». Et M. Cahn de préciser : « La tradition française, qui était de maintenir à distance les manifestants pour faire le moins de blessés, a évolué. Elle a progressivement laissé la place à une vision plus légaliste pour faire le moins de blessés, a évolué. Elle a progressivement laissé la place à une vision plus légaliste où les autorités vont moins rechercher le dialogue avec les syndicats au cours de la manifestation. les réponses apportées n'assurent pas l'équilibre fragile entre sécurité publique et libertés publiques. En effet, cette proposition de loi rogne clairement les libertés publiques, quoi qu'en disent ses défenseurs. Elle rogne notamment la liberté de manifester, nous laissant craindre la mise en place progressive des conditions permettant, à terme, de mettre fin à toute manifestation. Ridicule ! Comme l'a demandé mon collègue Pierre-Yves Collombat en commission, ne peut-on pas neutraliser quelques individus ultraviolents autrement qu'en violentant une fois encore les libertés publiques et en s'en prenant au code pénal ? Il est très inquiétant de constater que les articles 1 et 2 de la proposition de loi sont directement issus de la législation antiterroriste été aggravée l'année dernière, à la suite des nombreux renouvellements de l'état d'urgence et à l'instauration dans notre droit commun d'un certain nombre de dispositifs déployés dans ce cadre précis de menace terroriste. Le droit d'exception continue donc de polluer notre droit commun, au détriment des libertés individuelles et publiques ! Permettez-moi de rappeler que, en droit international, le droit à la liberté de réunion pacifique est inscrit dans les traités relatifs aux droits de l'homme auxquels la France est partie, comme les droits à la liberté d'association et à la liberté

remise, que, « eu égard à son économie générale, cette proposition de loi apparaît tout à la fois inutile et dangereuse et semble s'affranchir des exigences constitutionnelles et conventionnelles ». En droit En droit français, l'article X de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle, énonce clairement la liberté de manifestation des opinions : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi Ce ne sont pas les manifestants eux-mêmes qui troublent l'ordre public. En matière de sécurité publique, les forces de l'ordre n'ont sûrement pas besoin de ce genre de dispositif. En revanche, la rénovation de leurs moyens matériels et humains est urgente. L'explication de ces violences réside sans doute moins dans leur accroissement ou leur intensité hypothétiques que dans l'incapacité de nos forces de l'ordre à les démanteler et à remonter le fil de ces formations violentes, qui pourtant expriment bien souvent leurs intentions avant de frapper, faute de moyens suffisants. Mes chers collègues, il est grand temps de changer de paradigme, de cesser de s'inscrire dans le diptyque caricatural : tout-sécuritaire et répression ou tout-libertaire et laxisme !

elle n'est pas non plus anodine, parce qu'elle concerne les libertés fondamentales. En 1970, dans une société encore marquée par les événements de 1968, le gouvernement avait décidé de mettre à mal la liberté de manifester, au moyen d'une loi anti-casseurs qui provoqua de vifs débats.

cette accusation [ ...], selon laquelle, parce que nous critiquions votre projet de loi, nous étions les complices ou les défenseurs des casseurs. Cet argument est vil, cet argument est faux, cet argument est contraire à la tradition de notre parti et je tiens à vous dire que nous condamnons- je le proclame hautement

ne condamne que les manifestations issues des rangs de la gauche, sans critiquer les violences qui ont pu être observées dans les cortèges opposés au mariage pour tous lors du précédent quinquennat. Ce n'est pas correct on aperçoit sur des vidéos publiées par sur son site internet « des manifestants, certains cagoulés, s'en prendre aux forces de l'ordre, lancer des bouteilles, des barrières métalliques, des pavés ». Je rappelle également les pancartes et cris racistes parfois utilisés par certains manifestants des mêmes cortèges pour s'opposer à la garde des sceaux de l'époque, la courageuse Christiane Taubira. J'espère que mes collèguesde toutes les travées me rejoindront pour condamner cesdébordements.

soyez patient ! François Mitterrand, disais-je, s'opposa avec force à la loi anti-casseurs de 1970. Il déclara notamment : « En défendant son projet de loi, le gouvernement a voulu dire à l'opinion qu'il entendait frapper les commandos, les bandes organisées, les groupes qui agissent par la violence. S'il s'agissait de cela, on pourrait en discuter. Encore faudrait-il maintenir les garanties du droit ! Mais vous savez, les " formes nouvelles de la délinquance ", il n'y a rien de nouveau sous le soleil ! Et en réalité, nos lois, notre code pénal, permettent de répondre à cette question. « En vérité, le gouvernement a saisi l'occasion, comme s'il voulait profiter des circonstances, pour élargir incroyablement la délinquance possible. C'est ainsi qu'en fait il interdit désormais le droit de manifester, le droit de se réunir. Et beaucoup de gens, les parents des enfants mineurs, les organisateurs de réunions ayant l'intention d'être pacifiques, les organisateurs, les chefs, responsables, syndicalistes, politiques, les associations professionnelles, toutes tombent sous le coup de la loi. « Même dans des époques extrêmement rudes, au lendemain de la révolution de 1830, au lendemain des événements de 1934- les ligues, les ligues factieuses -ou de 1936, au moment où il y avait des conflits dans la rue, on n'est jamais allé si loin. Je ne veux pas croire, monsieur le président Retailleau, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs de la majorité sénatoriale, que vous souhaitiez vous inscrire dans l'héritage de cette triste loi de 1970. D'ailleurs, il me semble que M. Séguin et son groupe du RPR ne se sont pas opposés avec beaucoup de force à son abrogation. La raison en est simple : la loi de 1970 avait fait la preuve de sa dangerosité. Dans un éditorial du du 26 novembre 1981, Bertrand Le Gendre écrit : « Certes, les casseurs-ou prétendus tels -payèrent leur tribut à la loi nouvelle, mais aussi, très vite, des syndicalistes ouvriers, étudiants et paysans. Des procédures expéditives furent engagées contre les manifestants antinucléaires de Creys-Malville et de Plogoff. On vit même les musiciens anglais d'un groupe punk, les Stranglers, condamnés parce qu'un de leurs concerts avait dégénéré à Nice. Les critiques contre la loi anti-casseurs culminèrent après les incidents du 23 mars 1979 à Paris. Trente-cinq manifestants ou passants furent condamnés à la suite des violences commises place de l'Opéra. » C'est quoi, ça ? Wikipédia ? Certes, j'ai bien noté les amendements de Mme la rapporteur visant à rendre ce texte plus acceptable. Encore une fois, nous ne voulons pas donner l'impression d'esquiver le débat sur les dérives qui se produisent dans certaines manifestations. Mais nous craignons que le remède ne s'avère pire que le mal. Comme l'a rappelé Mme Troendlé en commission, « il serait erroné de dire que nous sommes, face à ces phénomènes de violence, complètement démunis ». Mais, à force de vouloir adapter le processus de maintien de l'ordre aux évolutions des casseurs, ne risque-t-on pas de mettre à mal la liberté de manifester ? Comme l'a rappelé notre collègue Thani Mohamed Soilihi en commission : « Les groupes qui sont visés font preuve d'ingéniosité : aussitôt repérés, ils inventent d'autres modalités d'intervention. Quand cette loi aura été adoptée, ils s'adapteront. Il vaut mieux faire porter l'effort sur le démantèlement de ces groupes.

Sont-ils devenus des citoyens de seconde zone ? Tous les supporters ultras ne sont pas des hooligans, comme tous les militants radicaux ne sont pas des casseurs. Je n'ai jamais dit cela ! Ce week-end, dans les stades de France, un quart d'heure de silence sans chant d'encouragement a été organisé pour protester contre la répression systématique dont s'estiment victimes les supporters. Dans la tribune de que je viens d'évoquer, ... De bonnes sources ! ... les auteurs déclarent : « Pour l'instant, il n'existe aucun dialogue ni aucune concertation, au point de faire des fumigènes un noeud de crispation répressif occultant d'autres problèmes réels dans les tribunes, comme le racisme, l'antisémitisme ou l'homophobie. On accuse et on condamne sans la moindre réflexion. Le recours punitif de plus en plus fréquent jusqu'au huis clos automatique, après des procès réalisés à la va-vite, au sein de commissions de disciplines partiales et sectaires, participe à l'envenimement des choses. » Ce constat m'inquiète. Doit-on manier davantage le bâton que la carotte, alors que l'ambiance des stades en France peut désormais rivaliser avec celles de nos voisins européens ? Le texte que nous examinons aujourd'hui, M. Grosdidier l'a relevé, s'inscrit dans cette philosophie. Il encourt les mêmes risques : décourager les manifestants comme on décourage les supporters. Mais non ! Au contraire ! On compte près de treize manifestations par jour à Paris. Comment pourrait-on techniquement émettre des interdictions ponctuelles dans cette ville ? Il existe, enfin, un autre risque démocratique majeur, celui de cibler certains membres d'organisations politiques et syndicales. Cette proposition de loi est à rebours de l'évolution actuelle. Sur le long terme, comme cela a déjà été dit, les historiens nous apprennent que les manifestations sont en réalité bien moins violentes que ne l'étaient les manifestations des XIX et XX siècles, comme on tend à l'oublier. Mais la tolérance à la violence, elle, s'atténue.

être attentif aux acteurs, aux slogans comme à leurs supports, et inscrire les manifestations dans le temps long de l'histoire sociale. On redécouvrirait alors l'inventivité de collectifs de graphistes producteurs de nouvelles images- gros succès, tout récent, du slogan-autocollant " Rêve-toi et Marx " -, la réapparition- encore timide -des chorales et des orchestres et, surtout, le syncrétisme de certaines luttes. » C'est un angle différent de celui qui a été retenu par les auteurs de cette proposition de loi, ... C'est sûr ! ... lesquels ont préféré se focaliser sur la violence. Il y a de la violence dans les manifestations. Il y en a toujours eu. Il s'agit de la contrôler et de l'éviter. Il ne s'agit pas d'éviter les manifestations. Ce n'est pas l'objectif ! Monsieur Retailleau, pour conclure mon propos, Monsieur Retailleau, pour conclure mon propos, je souhaitais vous poser une question sincère : que pensent les organisations syndicales, les partis politiques, les autorités judiciaires, les policiers et les militants associatifs de votre proposition de loi ? Et ? Et les voyous ? Vous n'avez sans doute pas réalisé d'étude d'impact, et je le comprends parfaitement. Mais avez-vous consulté dans un esprit de rassemblement ? Je vous pose cette question, non pas pour vous taquiner, mais pour vous aider à mener la réflexion sur la violence dans les manifestations que vous évoquez, je veux le croire, avec sincérité.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, madame la rapporteur, mes chers collègues, les événements du 6 février 1934 provoqués par des ligues nationalistes en face de la Chambre des députés, s'étaient soldés par 18 morts et plus de 3 000 blessés, dans un contexte économique, politique et organisationnel instable. Le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public est venu organiser le régime juridique des manifestations en instaurant un système de déclaration préalable à l'autorité administrative. D'autres mesures préventives telles que le renforcement du pouvoir de dissolution de groupes de combat et de milices privées ont rapidement été prises. En réponse aux événements de mai 1968, avec des affrontements d'une autre ampleur que ceux que nous connaissons aujourd'hui, la loi du 8 juin 1970 tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance, dite « loi anti-casseurs », a instauré une responsabilité pénale et collective des auteurs de violences. Jugée arbitraire, puisqu'elle permettait de condamner de simples participants à une manifestation qui n'avaient pas pris part aux actions, elle fut abrogée en 1981. Mes chers collègues, nous partageons la volonté des auteurs de la proposition de loi de lutter contre les violences lors des manifestations et de freiner le phénomène des Blacks Blocs, tant que nos libertés fondamentales demeurent préservées, parmi lesquelles la liberté d'aller et venir et le droit de manifester. Tout à fait ! Il est étonnant que la proposition de loi ne vienne pas illustrer par des chiffres la nécessité de légiférer pour renforcer un arsenal répressif en vigueur très complet, comme cela a été décrit par le rapport de la commission des lois. Alors que les formes de délinquance ne sont pas plus nouvelles ni plus violentes que celles que l'on a connues par le passé, il est proposé de restreindre davantage l'exercice de nos libertés individuelles. Cette proposition de loi, si elle part d'une intention louable, ne pouvait être adoptée en l'état, et je souhaite saluer le travail réalisé en commission par Mme la rapporteur, qui a tenté autant que possible de faire en sorte que ce texte ne sorte pas des bornes de la constitutionnalité. Je m'interroge sur l'inflation législative que nous connaissons, pour une efficacité contestable : nombreuses sont les mesures intégrées à cette proposition de loi qui sont satisfaites par notre droit en vigueur. le volet préventif de la proposition de loi, le contrôle des effets personnels des passants aux abords des manifestations est déjà existant. Une généralisation des contrôles, en élargissant le dispositif des périmètres de protection et de sécurité prévu pour l'état d'urgence, nous semble à la fois risquée sur le plan constitutionnel et impossible à mettre en oeuvre dans la pratique, au regard du nombre de personnes qui devraient être soumises à un contrôle. En ce qui concerne la possibilité pour le préfet de prononcer des interdictions administratives de manifester à l'encontre des individus susceptibles de représenter une menace pour l'ordre public, nous considérons que de telles interdictions doivent continuer d'intervenir dans un cadre judiciaire, plus protecteur des droits fondamentaux. En effet, il n'est pas souhaitable d'interdire de manifester des personnes qui n'ont jamais été condamnées pour des violences lors des manifestations, jugées sur leur simple comportement. À l'instar de l'article 3, qui prévoit la création d'un fichier national des personnes interdites de manifester, nous estimons que ces articles sont difficilement applicables. S'il est aisé de filtrer les entrées dans un lieu clos comme un stade, il s'avère très compliqué de bloquer l'accès à une manifestation en plein air. Il est donc préférable de maintenir le droit en vigueur, qui permet au juge de prononcer une peine complémentaire d'interdiction de manifester. Sur le volet répressif, l'article 4 vient ériger en délit la dissimulation volontaire du visage. Autant dire que cette disposition me paraît disproportionnée et d'une utilité limitée. Comme cela est clairement indiqué dans le rapport, la dissimulation du visage, actuellement sanctionnée par le code pénal, ne fait l'objet que d'un faible nombre de contraventions en temps normal. Lors d'une manifestation, les forces de l'ordre ont effectivement d'autres préoccupations. Encore une fois, le droit en vigueur reste plus judicieux en retenant la dissimulation du visage comme une circonstance aggravante. Enfin, le dispositif de responsabilité civile collective prévu initialement nous paraissait dangereux, parce qu'il laissait planer le risque qu'un individu puisse être accusé arbitrairement de dommages qu'il n'a pas causés. Cette mesure était disproportionnée et allait plus loin que la loi anti-casseurs- puisque le juge avait la possibilité de limiter la réparation à une partie des dommages et fixer la part imputable à chaque condamné en le dispensant de la solidarité.

Sur ces sujets, prenons le temps de la réflexion ! Le renforcement de l'arsenal juridique au cours de ces vingt dernières années n'a pas, pour le moment, fait ses preuves. Intégrons les conclusions de la commission d'enquête pour encadrer la présence d'intervenants extérieurs au sein des manifestations, ainsi que la réflexion conjointe menée par les ministères de la justice et de l'intérieur sur l'amélioration du traitement des infractions commises lors des manifestations. L'ensemble de ces éléments pourrait, je le pense, nous permettre d'avoir une vision plus complète du sujet afin, le cas échéant, de légiférer.

M. Stéphane Ravier. Monsieur le président, les frasques de M. Benalla ne doivent pas nous faire oublier que les manifestations autorisées et pourtant officiellement encadrées, tant par les organisateurs que par les services de police, sont devenues, depuis quelques années, l'occasion, pour essentiellement deux catégories d'individus, de se livrer à la plus extrême des violences : destruction de biens privés comme d'équipements publics allant même jusqu'à s'attaquer à un hôpital pour enfants ; agressions ultraviolentes envers les forces de l'ordre jusqu'à attenter à la vie de policiers en incendiant le véhicule dans lequel ils se trouvent Le poète a beau chanter que le rouge et le noir peuvent s'épouser, dans la rue, ils ne le font jamais pour le meilleur, mais ils le font uniquement pour commettre le pire ! Car les auteurs de ces actes insupportables, que professionnels, policiers, ou simples badauds subissent depuis des années sont principalement le fait des mouvances d'extrême gauche et d'anarchistes. Camouflées dans le treillis de l'antifascisme, qui, on le sait, permet au premier casseur ou clandestin venu d'extérioriser sa haine de tout ce qui peut représenter l'État, de tout ce qui peut représenter la France, ces milices utilisent les manifestations de masse pour les transformer en vastes opérations de casse. Ces derniers mois, ces groupes se sont servis de la loi Travail et des revendications légitimes des travailleurs pour tout détruire. Les uns sont issus du « ghetto » d'Auteuil-Neuilly-Passy, ces révolutionnaires de foire passant du cocktail au champagne au cocktail Molotov les autres, qui prétendent renverser la société, passent l'essentiel de leur temps à vivre à ses crochets. Les deux n'ont pas la notion du coût de ce qu'ils détruisent et ont en commun la haine de ceux qui nous protègent. Il y a quelques jours, ces fanatiques de la destruction, y compris de la démocratie, ont cassé une librairie en plein coeur de Paris, à quelques mètres du Sénat, sans que personne s'en soit indigné ! Le 28 avril, ce sont 24 policiers et gendarmes qui ont été blessés, dont 3 très grièvement à Paris. Le 14 juin, 29 policiers blessés. Le 15 septembre : 15 policiers blessés Comment ont-ils pu répéter leurs actes sans qu'aucune mesure ne soit prise ? Pourquoi a-t-on tant de complaisance pour cette racaille ? Pourquoi ne pointe-t-on pas leurs accointances avec les syndicats et les partis de gauche et d'extrême gauche ? Doit-on rappeler les débordements sans précédent, le 1 mai, de la part de plusieurs centaines de Black Blocks en plein coeur de la capitale ? Le prétendu antifascisme doit, lui aussi, avoir ses limites. Le climat d'impunité et l'absence totale d'État ne sont pas près d'être remis en cause par la nomination de Christophe Castaner au ministère de l'intérieur. En décembre 2015, celui qui battait encore pavillon socialiste en appelait à demi-mot à l'insurrection des quartiers en cas de victoire du Front national à l'occasion des élections régionales en Deux mesures suffiraient, si on les appliquait, à éradiquer cette violence. La première : dissoudre les milices d'extrême gauche et anarchistes ; ... et réactualiser, en y incluant l'expulsion du territoire national des casseurs étrangers, la loi dite « anti-casseurs » de 1970. Tout le reste ne serait que littérature et autant d'encouragements lancés aux casseurs pour perpétuer leur entreprise de saccage et d'agression de nos forces de l'ordre.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, madame le rapporteur, mes chers collègues, les violences dans les manifestations deviennent récurrentes CRS pris au milieu des flammes ; policiers blessés ou brûlés ; dégradations de bâtiments institutionnels, de mobilier urbain, de bâtiments commerciaux ; destructions d'équipements publicitaires ; voitures incendiées ; jets de projectiles contre les forces de l'ordre Ces faits font malheureusement trop souvent la « une » de l'actualité à l'occasion des manifestations. Les pouvoirs publics sont ainsi confrontés à l'émergence d'un phénomène nouveau, désigné par l'expression Black Blocs, qui fait obstacle à l'exercice de la liberté de manifester et remet en question la conception traditionnelle de l'ordre public. Ces individus veulent, par leur action violente, faire passer des messages politiques et exprimer leur haine de l'État et de toute forme d'autorité, ainsi que leur rejet de la mondialisation, du capitalisme et de la société de consommation. La radicalisation de l'action de ces groupes et mouvances contestataires lors des manifestations conduit à s'interroger aujourd'hui sur l'efficacité de l'arsenal juridique de maintien de l'ordre dont s'est doté notre pays au cours des dernières années. Le droit de manifester paisiblement, garanti par l'article X de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, semble aujourd'hui menacé en raison de ces actes violents de grande ampleur. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui prévoit notamment de rendre possible le contrôle des effets personnels des passants- contrôle visuel, ouverture des sacs et palpations de sécurité -lors des manifestations, lorsqu'il existe un risque de troubles à l'ordre public. Elle permet également de constituer, dans le respect des libertés publiques, un fichier de personnes interdites de manifestations et de créer un nouveau délit consistant à dissimuler son visage lors d'une manifestation sur la voie publique, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Elle prévoit aussi de considérer comme un délit, puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, lorsqu'il est commis lors d'une manifestation, le fait de détenir ou de faire usage, sans motif légitime, de fusées d'artifice ou de détenir toute arme par destination. Enfin, la proposition de loi rend l'ensemble des peines complémentaires prévues pour le délit de port d'arme lors d'une manifestation applicable à l'ensemble des infractions existantes ou nouvelles, en lien avec le fait de participer ou d'organiser ou d'organiser une manifestation et ajoute pour ces infractions la peine complémentaire d'interdiction de manifester. Le double volet, préventif et répressif, de cette proposition de loi a été approuvé et sécurisé par la commission des lois, grâce à l'adoption de dix amendements de son rapporteur, notre collègue Catherine Troendlé, afin de prévenir efficacement les atteintes à l'ordre public, dans le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis. Dans le cadre du volet préventif, les préfets pourraient faire contrôler les effets personnels des passants dans le périmètre et aux abords immédiats d'une manifestation. Ils pourraient aussi prononcer, à l'encontre des individus susceptibles de représenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, des interdictions personnelles de manifester, assorties le cas échéant d'une obligation de pointage dans un commissariat ou une gendarmerie. La création d'un fichier national des personnes interdites de prendre part à des manifestations serait également prévue. Dans le cadre du volet répressif, l'infraction de dissimulation volontaire du visage dans une manifestation, dans des circonstances faisant craindre des troubles à l'ordre public, actuellement punie d'une contravention de la cinquième classe, serait transformée en un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'infraction de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme serait étendue afin de viser aussi les abords immédiats de la manifestation et de sanctionner la tentative de ces délits. Le champ de la peine complémentaire d'interdiction de manifester serait par ailleurs élargi. Par ailleurs, la proposition de loi, dans sa rédaction initiale, prévoyait d'instaurer une présomption de responsabilité civile collective en matière de dommages causés à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique. La commission des lois a préféré maintenir le régime de responsabilité sans faute de l'État, tout en offrant à celui-ci la possibilité d'exercer une action récursoire contre les personnes condamnées pour les violences ou dégradations à l'origine de ces dommages. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants votera ce texte ainsi modifié et enrichi par notre commission des lois.

il y a quelques mois, des violences d'une gravité inadmissible ont eu lieu en plein Paris. Des commerces ont été détruits. Des personnes auraient pu mourir, si elles n'étaient pas parties à temps. La préfecture de police était confrontée non pas à des manifestants qui exercent leur droit de manifester, mais bien à des casseurs, à des gens sans foi ni loi, qui veulent détruire et même tuer. Ils n'ont que de la haine pour les forces de l'ordre et de la haine pour la société. Ces casseurs profitent des faiblesses de notre législation. Leur envie est d'autant plus aiguisée qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. Ils testent notre réactivité en jouant sur nos propres limites. Cette situation est anormale. Il est choquant que des individus profitent des faiblesses de l'État de droit pour commettre leurs délits. C'est à cette lacune que cette proposition de loi, due à l'initiative de Bruno Retailleau, entend remédier. Il n'y a pas de violation des libertés publiques quand on cherche à sévir contre ceux qui veulent casser, tuer ou mettre en danger la vie d'autrui. Ceux qui détruisent les commerces de cette France qui travaille, de cette France qui se lève tôt ne méritent pas la protection de la Nation. Ils doivent être mis hors d'état de nuire. Ils doivent être pris pour ce qu'ils sont : des délinquants, voire des criminels. Manifester est un droit, c'est le droit d'exprimer une opinion ; il est parfaitement légitime. La République ne prétend pas régir les consciences. Chaque citoyen a droit au désaccord et au dissentiment. Il a le droit de le faire savoir. C'est la règle du jeu dans tout État démocratique. Mais dans tout État de droit, il y a une contrepartie, une responsabilité à respecter. Ainsi, la République se doit d'exiger que l'on manifeste à visage découvert. Je comprends mal cette envie d'anonymat de la part de ceux qui se masquent intégralement ... ou plutôt je comprends trop bien qu'il s'agit là d'une lâcheté qui s'ajoute à leur violence. Après tout, une manifestation est un acte public, où l'on assume son opinion ouvertement et sans détour. Il est incompréhensible que certains profitent de cette occasion pour dissimuler leurs sombres desseins. Pour cette raison, je soutiens fortement la création d'un nouveau délit visant à punir la dissimulation du visage lors de manifestations et de rassemblements. Cette non-dissimulation est une exigence de bon sens. Il ne s'agit plus de porter atteinte à la vie privée, puisqu'une manifestation est un acte qui se déroule dans l'espace public.

Depuis lors, personne ne songe à y revenir. Oui, la République ne se vit pas cachée. Évidemment, le dispositif envisagé dans cette proposition de loi n'est « pas applicable aux manifestations conformes aux usages locaux C'est en effet ce que prévoit le projet d'article du code pénal. Nous voulons sévir contre les Black Blocs, pas contre Belphégor ! On peut parfaitement distinguer le respect d'une tradition des débordements À l'occasion de sa prochaine évasion, Rédoine Faïd n'aura plus besoin d'une burqa, mais il se mêlera aux Black Blocs pour se dissimuler à nouveau ... N'attendons donc pas ! De même, il faut améliorer nos dispositifs concernant la responsabilité des dégradations commises collectivement. Entendons-nous bien : il s'agit non pas de sanctionner des personnes qui n'ont rien fait, mais de sévir contre celles qui sont responsables d'actes violents et qui ont été condamnées en conséquence. Il s'agit de permettre à l'État de se retourner, par une action récursoire, contre ceux qui ont été condamnés pénalement pour violence contre les personnes ou atteintes aux biens. Il est normal que ces personnes aient à répondre des dommages résultant de la manifestation elles ont profité de cette manifestation pour casser et mettre en danger la vie d'autrui ; elles doivent donc en assumer les conséquences et réparer les dommages commis. Mes chers collègues, il y a urgence en la matière, notamment à Paris, mais aussi en province. Je pense en particulier aux événements qui se sont déroulés à Nantes dont a parlé Bruno Retailleau. Et à Rennes ! Et je salue tous mes collègues élus de grandes villes qui subissent ces violences inadmissibles. Nous n'en pouvons plus de ces rassemblements qui dégénèrent. N'attendons pas le pire ! Les violences urbaines sont inexcusables. Pour toutes ces raisons, en accord avec mes collègues du groupe Les Républicains, qui ont porté ce texte, je voterai cette proposition de loi, et j'invite tous les sénateurs à voter ce texte qui doit emporter l'adhésion la plus large. Je demande au Gouvernement et au professionnel que vous êtes, monsieur le secrétaire d'État, d'entendre la voix de ceux qui n'en peuvent plus de cette impunité récurrente des casseurs. La parole

En effet, le code pénal reconnaît et protège ces libertés. Il punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de de réunion ou de manifestation. Si nous comprenons parfaitement que les participants à une manifestation puissent afficher une certaine forme de véhémence- véhémence des propos tenus par les leaders syndicaux, véhémence dans les mots d'ordre de la manifestation aucune violence ni aucune atteinte aux personnes et aux biens ne peuvent être tolérées. Au-delà de prévenir et de sanctionner les violences, l'enjeu de cette proposition de loi, mes chers collègues, est donc bien de protéger la liberté d'expression. Certains de nos concitoyens ne vont plus manifester, car ils ont peur. Ils se sentent de plus en plus souvent en insécurité dans l'espace public lors des manifestations. Le droit de manifester, corollaire de la liberté d'expression, est en train de s'user en raison de ces violences aujourd'hui récurrentes de groupes organisés. Nous ne pouvons l'accepter Ces groupes organisés, dénommés Black Blocs, se joignent aux manifestants, non pas pour revendiquer des droits ou défendre leur profession, mais exclusivement pour casser : casser du mobilier public, casser des biens privés, tels que des vitrines, mais aussi « casser du flic » et piller les magasins, ce qui donne lieu à de véritables scènes d'émeutes urbaines. En dissimulant leurs visages avec des foulards, des cagoules ou des casques, les membres de ces groupes contreviennent à la législation en vigueur, qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Ils démontrent surtout leurs intentions belliqueuses. Ces comportements violents font reculer la liberté d'expression. La proposition de loi sur laquelle nous allons débattre permettra non seulement des manifestations, mais aussi de donner les moyens légaux à la police d'appréhender les causeurs de trouble, et à la justice de les condamner puis de les tenir à l'écart des futurs rassemblements. Ainsi, la création d'un fichier de personnes condamnées à la peine d'interdiction de participer à des manifestations, dans le respect des libertés publiques, est un outil indispensable pour éviter que les violences ne se reproduisent. De même, l'interdiction préalable de prendre part à une manifestation ou la convocation au commissariat de police au moment de la manifestation, en cas de risque d'une particulière gravité pour l'ordre public, sont des mesures qui ont déjà fait leurs preuves- je suis d'accord à ce sujet notamment dans les stades de football. Nul doute que ces dispositions permettront aussi de pacifier les manifestations sur la voie publique et qu'elles garantiront ainsi à nos concitoyens un usage serein de leur droit de manifester. En tant que législateurs, mes chers collègues, il est de notre devoir de garantir à chacun de nos concitoyens le droit de manifester paisiblement et en sécurité dans l'espace public. Ce droit, cette liberté de se réunir et de manifester sur la voie publique accordée à chaque Français, est remise en cause par la violence de ces groupes organisés, prêts à en découdre avec l'ordre public républicain. Dans le respect des libertés publiques, il nous appartient de protéger un des droits fondamentaux garantis par l'article X de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celui de pouvoir s'assembler

On espère ici que vous l'insufflerez à votre ministre de tutelle qui, la semaine dernière, a été particulièrement désagréable à l'encontre de notre collègue Philippe Dallier lors des questions d'actualité Nous aurions pu penser qu'avec un arsenal juridique étendu, complet, voire complexe, et même renforcé ces dernières années, la France était en mesure de répondre à toutes les situations impliquant des opérations de maintien de l'ordre. Force est de constater que de nouveaux phénomènes violents et de nouvelles menaces à l'ordre public nous obligent aujourd'hui à légiférer et à compléter nos moyens d'action, tout en garantissant les libertés fondamentales, comme le droit de manifester. Manifester, c'est protester ; ce n'est pas casser, ni blesser, ou intimider. Toutes celles et ceux qui pensent que la violence peut se légitimer par des motifs politiques sauront que l'État de droit doit être respecté en tout temps et en tout lieu. Ces dernières années, l'ouest de la France a été le théâtre de nombreuses exactions et d'actes de vandalisme autour de l'emblématique dossier de Notre-Dame-des-Landes, qui est aussi un emblématique fiasco du gouvernement actuel, et un renoncement du Président de la République à sa promesse de campagne.

Les centres-villes de Nantes et de Rennes ont souvent été vandalisés ces dernières années, les équipements publics détruits, les vitrines brisées par des groupuscules ultraviolents. L'année 2014 a été localement marquée par la grande manifestation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, une des manifestations les plus violentes dans l'histoire de Nantes, même s'il n'y eut heureusement aucune victime. Toujours à Nantes, en 2016, plus d'une centaine de policiers ont été blessés lors des manifestations contre la loi Travail. du mois d'avril 2016, il est fait mention d'un groupe de 600 casseurs au profil particulièrement hostile. Encore à Nantes, le 22 mars 2018, des heurts violents ont éclaté entre un groupe de manifestants anticapitalistes, visage dissimulé, et la police. enfin, le 19 avril dernier, une centaine d'individus cagoulés ont harcelé les forces de l'ordre. On a recensé à cette occasion de multiples dégradations. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle reflète la répétition des actes violents. Ces épisodes sont inadmissibles dans un État de droit. Le taux des individus interpellés qui ont été déférés à la justice est faible. Je tiens à saluer le travail exceptionnel et le calme des forces de l'ordre, dont la tâche n'est pas des plus simples dans un contexte de plus en plus dégradé. Ce texte a le mérite de compléter notre arsenal juridique de façon concrète, parce qu'il est souvent difficile de déterminer les responsabilités et de rassembler les preuves dans le désordre des mouvements de masse. Les dispositions proposées aujourd'hui seront également utiles aux préfets, dont la connaissance du terrain permet d'adapter les dispositifs et de graduer la réponse selon les circonstances propres à chaque manifestation. Enfin, il serait utile pour l'État de pouvoir se retourner contre les casseurs pour s'assurer qu'ils participent à l'indemnisation des victimes. Quand on observe l'ampleur des dégâts à Nantes et à Rennes après ces manifestations, il faut bien reconnaître que le principe La résilience d'une nation se mesure aussi à sa capacité d'absorber de tels soubresauts avant que leur multiplication ne devienne incontrôlable. Je vous invite à y réfléchir durant le débat et, pour ma part, je soutiendrai cette proposition de loi de bon sens et, surtout, de responsabilité !

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, chacun d'entre nous garde en mémoire les violences et les dégradations qui ont émaillé toutes les grandes manifestations récentes, notamment celle du 1mai à Paris. Les atteintes aux biens sont naturellement inacceptables, mais les atteintes aux personnes le sont encore plus, lorsqu'il s'agit de policiers ou de gendarmes. De tels saccages et agressions ne sont pas nouveaux. Certes, mais comment s'en satisfaire ? Sommes-nous condamnés au fil des ans à être les spectateurs de ces scènes de guérilla, de ces commerces incendiés, de ces CRS blessés ? Certainement pas ! Il faut utiliser tous les moyens pour que chacun puisse continuer à exercer son droit de manifester dans notre pays. Une manifestation ne saurait créer une zone de non-droit dans laquelle on peut se livrer à toutes les exactions, à toutes les violences, en se sentant protégé par une foule anonyme. Pour mettre un terme à ces dérives, les moyens que l'on peut utiliser sont d'abord matériels s'assurer que nos forces de sécurité soient parfaitement équipées, aussi bien pour se protéger que pour détecter et faire cesser efficacement un rassemblement qui bascule dans la violence. Ensuite, il faut des moyens juridiques pour poursuivre efficacement les individus violents qui se croient intouchables, parce que masqués et noyés dans la foule. Les auteurs de la présente proposition de loi visent ici un objectif bien précis, qui appelle une évolution de notre droit. Le phénomène dit des Black Blocs s'est développé récemment. Le 1mai dernier, à Paris, ils étaient près de 1 200. À titre de comparaison, en 2016, ils étaient 200 ; en 2017, environ 800. La tendance est donc assez nette. se trouvent démunis pour poursuivre ces délinquants utilisant des techniques de dissimulation élaborées et concertées. Dans les manifestations, les Black Blocs forment des groupes éphémères, dont l'objectif est de commettre des actions illégales, en formant une foule anonyme non identifiable. Ces individus portent des vêtements noirs ou très sombres, et dissimulent leur visage, ce qui rend difficile le travail d'identification et d'interpellation. Ils s'habillent ainsi au dernier moment et changent immédiatement de tenue une fois les exactions terminées. Voilà pour le constat. Comme l'a rappelé notre rapporteur, le dispositif figurant dans la proposition de loi a deux volets : l'un préventif, l'autre répressif. Nous partageons cette démarche globale consistant à donner de nouveaux instruments à l'autorité administrative avec, par exemple, les fouilles préventives, et à créer des dispositions pénales qui tendent à sanctionner plus sévèrement les auteurs de violences et de dégradations dans les manifestations.

Cette infraction existe depuis 2009, mais il s'agit de lui donner une tout autre portée, puisque le texte fait de cette simple contravention un délit passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

qui a pour objet d'autoriser la création d'un traitement de données à caractère personnel destiné à répertorier les mesures d'interdiction individuelle de manifester. Il s'agit, autrement dit, d'un nouveau fichier de police. Dans sa version initiale, cette disposition pouvait susciter quelques craintes, car elle retenait une définition très large, voire trop large, des finalités de ce fichier, et semblait disproportionnée au regard de de l'objectif à atteindre. Grâce au travail de notre rapporteur, dont je veux ici saluer la qualité, le texte issu des travaux de la commission des lois corrige ce défaut en limitant les finalités du fichier et en prévoyant que le décret en Conseil d'État, prévu en l'application de l'article, sera pris après publication d'un avis motivé

pour l'ensemble du texte, une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. Nous saluons ainsi les modifications introduites en commission, qui apportent un certain nombre de garanties supplémentaires. Ne soyons pas naïfs, cette proposition de loi ne permettra pas d'éradiquer toutes les formes de violence lors de manifestations. elle permet de mettre hors d'état de nuire les individus les plus violents et dangereux. Si elle permet de limiter les dégradations ou les agressions dont sont victimes policiers et gendarmes chargés d'assurer le maintien de l'ordre, alors, oui, elle est utile Convaincus que cette proposition de loi n'est ni une atteinte insupportable à la liberté de manifester ni une loi inapplicable, comme certains collègues l'ont affirmé en commission, les membres du groupe Union centriste la voteront ! La parole

les policiers travaillent sous une contrainte qui est extrêmement forte en matière d'ordre public. Comme vous le savez, ils tombent sous le coup de la loi comme tout et sont soumis à un contrôle très précis de l'Inspection générale de la police nationale, notamment. Je voudrais également rappeler que la qualification de violence policière ou d'usage excessif de la force

lorsque le texte a été consolidé par la commission des lois. Je les ai conviés à un petit-déjeuner de travail pour qu'ils m'expliquent quelles étaient leurs inquiétudes et que je puisse, de mon côté, leur expliquer quelle était la démarche de la commission des lois. Cet échange

à la lecture de cette proposition de loi, je ne peux qu'approuver les mesures visant à empêcher l'irruption d'individus violents dans les manifestations en favorisant leur interpellation et plus encore leur condamnation. J'approuve particulièrement ce texte dans son volet préventif, qui rend possible le contrôle administratif des effets personnels des passants lors des manifestations, dès lors qu'existe un risque de trouble à l'ordre public. Je l'approuve également, au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois lors de manifestations où des centaines de Black Blocs encagoulés, issus de la mouvance radicale d'extrême gauche, ont fait irruption au cri de « Tout le monde déteste la police » et ont gravement menacé l'ordre public, perturbant au passage le traditionnel défilé organisé dans le cadre de la fête du travail. On peut toujours s'interroger sur la nature composite de cette nouvelle forme de contestation violente et des références politiques qui s'y attachent : une part d'anarchisme, de marxisme, de situationnisme, des anciens autonomes, une frange libertaire et même une curiosité, des « animalistes », figurez-vous, qui auraient cassé le McDonald's lors des manifestations du 1 mai. Il faut dire que les bouchers sont désormais bien placés pour savoir que ces militants ne sont pas toujours très pacifiques ... Bien que ce phénomène soit parfois difficile à identifier, il n'en demeure pas moins que le législateur ne peut se contenter d'observer, d'analyser ou même de commenter, comme l'ancien ministre de l'intérieur Gérard Collomb, qui avait

et appelé les manifestants à « ne pas être complices de ce qui se passe par leur passivité ». Il s'agissait là d'une réponse très baroque et même dérisoire face à l'impuissance de l'État, attaqué comme tel, incapable d'interpeller et de faire condamner les auteurs de violences. qu'une partie de ces groupes s'est retrouvée dans les blocages des universités, voire des lycées, il y a quelques semaines, ou encore lors d'une manifestation autoproclamée « antifasciste » et dite « festive », organisée le 22 septembre dernier dans les rues d'Angers. il y a là une forme de nihilisme qui menace l'ordre public et, particulièrement, nos forces de l'ordre, cible revendiquée et particulièrement exposée. L'État doit donc réagir et mobiliser tous les moyens nécessaires pour sanctionner ces apôtres de la violence pour la violence

le sérieux et la rigueur intellectuelle de la commission des lois pour y avoir siégé pendant de longues années. Toutefois, je pense qu'il aurait été intéressant pour la bonne tenue de nos travaux de préciser,

L'article 1 confère aux préfets des pouvoirs disproportionnés en matière de sécurité publique. Les mesures ici adaptées au cadre particulier des manifestations risquent en outre d'en favoriser une application discriminatoire, dès lors que les fouilles ne requièrent aucune base objective. Sur quels critères s'opéreront les contrôles visuels et les palpations de sécurité, alors que la problématique bien réelle des contrôles au faciès, par exemple, reste aujourd'hui sans réponse de la part des gouvernants successifs de notre

Benbassa, sur l'article. Le présent article vise à instaurer un contrôle des effets personnels des passants lors des manifestations. Il s'agit d'une mesure conditionnée à l'existence de troubles à l'ordre public. Cet article prévoit également la mobilisation des agents de la police judiciaire chargés de procéder aux contrôles administratifs. Cette mesure coercitive, en plus de conférer un pouvoir arbitraire aux forces de l'ordre, est contraire aux libertés fondamentales. Ce contrôle est de surcroît impraticable et populiste : impraticable, car l'examen d'un rassemblement de 25 000 personnes, par exemple, durerait des heures

afin, directement ou indirectement, d'étouffer ou de décourager des mouvements de protestation ». Mes chers collègues, on se sert

dans la rue. Le contrôle des foules est un procédé liberticide. Si nous ne nous opposons pas à une telle mesure répressive, la France pourrait subir une énième condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que le droit de manifester est consubstantiel à l'exercice d'une citoyenneté et d'une société démocratique en bonne santé, nous ne saurions tolérer l'autoritarisme et la répression des cortèges ! Je suis saisi

la présente mesure est déjà encadrée par le droit et appliquée sur le terrain. Le droit permet d'ores et déjà la mise en place d'un dispositif de filtrage des manifestants. Ce dispositif figure parmi un ensemble de mesures préparatoires, qui ont lieu en amont de la manifestation, et peut être mis en oeuvre sur le site et aux abords du site. Il vise à détecter les individus interdits de manifestation et et à limiter les risques de détention d'armes. Ensuite, il nous semble que la judiciarisation du maintien de l'ordre fournit aux forces de l'ordre un cadre juridique sécurisant au niveau procédural. On sait que les réquisitions sont généralement délivrées la veille pour des lieux et des périodes déterminés. Enfin, le présent un caractère disproportionné, car celui-ci tend à introduire dans le droit commun un recours au dispositif des périmètres de protection et de sécurité de l'état d'urgence, prévu à l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure. Si le Conseil constitutionnel reconnaît un caractère spécifique lié à la menace terroriste justifiant des atteintes fortes aux droits et libertés individuels, il ne saurait en être de même avec la prévention des actes délictuels commis

identiques visent à supprimer l'article 1 et sont par conséquent contraires à la position de la commission des lois. Cette dernière considère que la mise en oeuvre des périmètres de contrôle aux abords d'une manifestation présente un certain intérêt dans la mesure où elle permettra, grâce au filtrage des passants, de mieux sécuriser les manifestations. En raison des risques d'inconstitutionnalité que présentait le texte initial, la commission a complété l'article 1 de plusieurs garanties que je vais énumérer. Il y a d'abord l'encadrement dans le temps et l'espace des périmètres de contrôle, qui ne pourront désormais être instaurés que six heures au lieu de douze heures avant la manifestation. Ensuite, nous avons veillé à adapter les mesures de contrôle pour les personnes résidant ou travaillant dans le périmètre. Enfin, la commission a supprimé- j'y reviendrai plus tard -l'intervention des agents de police municipale et des agents de sécurité privée dans ces périmètres. Grâce à ces modifications, mes chers collègues, nous avons abouti- j'en suis personnellement convaincue -à un texte équilibré, qui écarte toute atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement

Le groupe de travail mis en place par le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice, visant à mieux détecter, interpeller et sanctionner les fauteurs de trouble lors des manifestations, constitue le cadre idéal pour cette réflexion. Il rendra ses conclusions au mois de janvier de l'année prochaine. Le Gouvernement est néanmoins défavorable à ces amendements de suppression.

de représenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, une interdiction de manifester, assortie, le cas échéant, d'une obligation de « pointage » auprès d'un représentant de l'autorité publique.

à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics Autrement appelé « interdiction de séjour prononcée en vertu de l'état d'urgence », ce dispositif avait été censuré par le Conseil constitutionnel, puis réécrit pour être réintroduit dans la loi, avec des garanties contre les atteintes à la vie privée et familiale des personnes visées par la mesure. Il est intéressant de noter que la rapporteur a introduit les mêmes modifications pour contourner le caractère anticonstitutionnel de la mesure initiale. Pourtant, comme Éliane Assassi l'indiquait dans son intervention générale,

L'amendement que nous présentons à cet article 2, défendu par cette intervention, vise à s'opposer à la transposition de la législation antiterroriste pour l'encadrement des manifestations. La disproportion des mesures de police administrative choisies ne permet pas d'assurer un équilibre entre maintien de l'ordre public et respect du droit constitutionnel de manifester.

en créant des contrôles administratifs systématiques à l'abord des manifestations et en favorisant des interdictions de manifester personnelles sans en définir les critères ni prévoir de recours effectifs et, d'autre part, à s'affranchir des exigences légales en matière de preuve.

présenter l'amendement n° 3. Nous avons bien compris que l'article 2 de la proposition de loi tend à créer une interdiction administrative individuelle, et non générale, de manifester. Trois raisons ont motivé le dépôt de cet amendement de suppression. point, il nous semble que la faculté de prononcer une interdiction de manifester existe déjà dans notre droit. Elle s'applique au moyen du recours à une peine complémentaire pouvant être prononcée par le juge pénal, peine complémentaire prévue par l'article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure. Deuxième point, notre attention a été l'aspect opérationnel de cette mesure. Dans la pratique, la mise en oeuvre d'une telle disposition nous semble très compliquée. Une mesure de cet ordre se traduirait par une charge de travail supplémentaire pour les forces de police, surtout si l'interdiction vise quantité de personnes. En outre,

Enfin, il nous semble qu'il faut faire confiance aux forces de l'ordre dans l'application de nouvelles techniques de désescalade face aux émeutiers. Là encore, on en revient à la doctrine d'emploi des forces de l'ordre. Troisième et dernier point, comme pour l'article 1, la mesure préconisée est disproportionnée. Elle conduit, de fait, à transposer dans le droit commun l'interdiction administrative de séjour de l'état d'urgence, en la concentrant sur les manifestations se déroulant sur la voie publique.

compléterait utilement le champ des prérogatives aux mains de l'autorité préfectorale pour prévenir les débordements à l'occasion d'une manifestation. De même que l'interdiction de stade, dont elle s'inspire d'ailleurs, cette mesure permettra d'écarter, avant même le début de la manifestation, les individus animés par la seule volonté de commettre des dégradations. Il s'agit de garantir l'exercice de la liberté de manifester pour les manifestants pacifiques.

elle a également encadré l'étendue géographique de l'interdiction de manifester. Troisièmement, elle a introduit une obligation de notification de l'interdiction à l'intéressé, afin de lui permettre de saisir, le cas échéant, le juge des référés. Il s'agit de garantir un droit au recours effectif. Grâce à ces apports, la commission des lois est parvenue à un texte utile,

effectivement 106 fichiers qui sont mis à la disposition des forces de sécurité, et encore, c'est sans compter les fichiers utilisés ou gérés par la préfecture de police de Paris. L'article 3 est d'autant plus inutile, selon nous, que les personnes condamnées à une peine complémentaire d'interdiction de manifester font déjà

n° 11 rectifié. L'article 3 de la proposition de loi faisant, aujourd'hui, l'objet de nos débats tend à la création d'un fichier de personnes interdites de manifestation. Avec cette mesure, deux écueils se présentent à nous. se pose la question du fichage. Au regard de l'histoire de notre Nation, ce procédé ne vous interpelle-t-il pas, mes chers collègues ?

Le régime de Vichy n'a-t-il pas été précurseur en matière de création de registres dès 1940, avec, notamment, le fameux « fichier Tulard », constitué par la préfecture de police de Paris ? Nous Pour cela, et à raison, le Conseil constitutionnel a toujours été réticent à la mise en place de tels listings. C'est insupportable ! En atteste notamment sa décision du 22 mars 2012

Cet article pose ensuite le principe de la restriction du droit à manifester. Ce droit, en France, n'est certes pas constitutionnel, mais il est protégé par l'article X de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, découlant du principe de la libre manifestation des opinions. Il ne s'agit pas du droit de casser ! S'il a pu être encadré par le passé, notamment en 1934 à la suite des manifestations de l'Action française, les actuelles protestations de l'opposition de gauche contre la politique antisociale du Gouvernement ne sauraient être assimilées au péril fasciste d'antan. Cela va de soi. Cet article est non seulement attentatoire au respect de la vie personnelle

par l'article 34 de la Constitution, au domaine de la loi. Ce n'est en fait qu'à raison de l'enregistrement de condamnations pénales- ici la peine complémentaire d'interdiction de manifester prévue par le code de la sécurité intérieure -et si le fichier est mis en oeuvre par un service autre que le ministère de la justice qu'une autorisation par la loi serait nécessaire, en application de l'article 777-3 du code de procédure pénale. La commission des lois ayant ajouté le ministère de la justice en tant que responsable du traitement, en supplément du ministère de l'intérieur, l'intervention d'une disposition législative ne semble plus nécessaire.

lorsque vous assimilez la proposition de la commission des lois aux

pour la sécurité nationale ! Quand une république comme la République française se défend, dans le respect du droit, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, en mettant en oeuvre de nouvelles législations destinées à empêcher les casseurs de venir disqualifier un certain nombre de manifestations pacifiques et de porter atteinte aux biens de contribuables français, d'honnêtes citoyens, je dois vous le dire, je ne me sens ni fasciste,

Voilà dix ans, Nicolas Sarkozy proposait le fichage de personnes atteintes de pathologies mentales hospitalisées d'office. Si le Président de la République de l'époque a reculé, le procédé semble toutefois s'être popularisé

visés par ce procédé démagogique et populiste. Non, les casseurs ! Par cette mesure, visant à interdire de manière préventive la présence de certains militants à des rassemblements ... Des

préventive la présence de certains militants à des rassemblements, une atteinte de poids est portée à l'article IX de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, portant sur la présomption d'innocence. Ainsi, nous ne pouvons que saluer

Néanmoins, ces avancées ne sauraient rendre ce texte acceptable. La commission, afin de se conformer à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a demandé que la confection d'un tel fichier se fasse après avis de la CNIL. Une telle solution nous paraît bien faible au regard des enjeux. C'est pourquoi nous proposons d'encadrer davantage encore le fichage des manifestants, en plaçant celui-ci sous un contrôle strict par la CNIL, en coopération avec la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la

qui serait exercé par la CNIL et la CNCTR. En application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le fichier prévu à l'article 3 de la proposition de loi sera effectivement soumis, comme tous les traitements de données à caractère personnel, à un contrôle de la CNIL. Introduire dans la loi un nouveau fondement juridique pour le contrôle serait source de confusion. Je propose donc que l'on en reste au droit actuel, donc à ce contrôle par la CNIL. Esther Benbassa propose également une participation de la CNCTR à ce contrôle. Pour avoir été membre de cette instance, je puis vous affirmer, mes chers collègues, qu'elle n'est

sur l'article. Cet article tend à sanctionner plus sévèrement les auteurs de violences et de dégradations dans les manifestations, en faisant de l'infraction de dissimulation volontaire du visage dans une manifestation dans des circonstances faisant craindre des troubles à à l'ordre public un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cette infraction est actuellement punie d'une contravention de la cinquième classe. Selon nous, en continuant d'aggraver les sanctions, les auteurs de ce dispositif continuent à traiter les causes, non les symptômes. Modifier l'échelle des peines au gré des fins politiques ne mènera jamais à la résolution des problèmes. Nous sommes là dans la pure illustration de l'échec de la répression. les auteurs de cette proposition de loi continuent à se fourvoyer, même si aucune infraction nouvelle n'est créée, les comportements visés étant déjà constitutifs d'infractions pénales- violence, dégradation et destruction de biens, port d'armes ... Au lieu de renforcer des sanctions qui existent déjà, donnons plutôt aux forces de l'ordre les moyens de démasquer en amont les individus. Or l'état de déshérence dans lequel sont plongées les forces de l'ordre les empêche de remonter le fil des organisations violentes qui, pourtant, annoncent bien souvent leurs intentions avant d'agir. À cet égard, il semblerait que les groupuscules ayant frappé lors de la manifestation du 1 mai dernier aient annoncé leur « mobilisation » sur les réseaux sociaux, au moins la veille des troubles visés.

si manifester n'est pas mon mode d'expression habituel, je me battrai toujours pour la liberté de manifester. Il faut pouvoir manifester en toute sécurité et cet article,

parce que les forces de l'ordre peuvent être amenées à contrôler par des moyens un petit peu durs ces individus et qu'il peut y avoir des victimes collatérales

le droit en vigueur admet aujourd'hui deux cas d'interdiction de dissimulation du visage. D'une part, l'article R. 645-14 du code pénal punit d'une amende de 1 500 euros « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public », hormis le cas où les manifestations sont conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. légitime. D'autre part, l'article 3 de la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public fait de la dissimulation du visage une circonstance aggravante de certaines infractions. L'article 431-4 du code pénal issu de la loi précitée fait ainsi de la dissimulation du visage une circonstance aggravante du délit consistant à « continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations Ainsi, l'interpellation n'est possible que lorsque la dissimulation du visage s'accompagne de la commission d'un délit ou de la tentative de commettre un délit, exigence qui permet de consolider la procédure, puisqu'il faut apporter une double preuve que le contrevenant masqué se dissimule le visage afin de ne pas être identifié, de manière volontaire ; en second lieu, qu'il existe des « circonstances de nature à faire craindre des atteintes à l'ordre public ». Dès lors, on peut considérer que la création d'un tel délit est inutile, voire disproportionnée, pour lutter contre la délinquance, car, si elle est censée faciliter l'interpellation et le placement en garde à vue, en pratique, elle ne rendra pas plus aisé le fait d'aller chercher les individus cagoulés au coeur d'une manifestation.

Je rappelle que l'article 4 vise à créer un délit de dissimulation du visage dans une manifestation dans le but de ne pas être identifié par les forces de l'ordre dans des circonstances faisant craindre un trouble à l'ordre public.

que la sanction prévue par la proposition de loi pourrait être plus dissuasive que l'actuelle contravention dont, faut-il le rappeler, le plafond est de 1 500 euros. Si elle devient

article tend à élargir l'infraction de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme, afin de viser non seulement le port d'arme, mais aussi le port d'arme par destination et celui de de fusées et d'artifices. Je suis au regret de constater que sont clairement visés, à travers cet article, non pas les Black Blocs, mais bien certains syndicalistes. Je pense en particulier aux cheminots ou aux dockers, qui peuvent utiliser de manière pacifique ce genre d'artifices, non pour en faire usage d'arme, mais bien plutôt pour marquer leur colère dans l'espace public, se faire entendre et se faire voir. Tel est l'objet des manifestations revendicatives, me semble-t-il. En outre, nous nous interrogeons sur la notion d'arme par destination et ce qu'elle pourrait englober. La latitude que se laissent les auteurs de ce dispositif est en cela particulièrement inquiétante et nous laisse pour le moins songeurs quant à leurs intentions réelles. J'ai J'ai un doute : ne s'agit-il pas tout bonnement de mettre en place les conditions pour censurer finalement toute forme de manifestation dans l'espace public ?

L'ONG chrétienne alerte les autorités françaises sur la dangerosité des armes dont elles se dotent et sur le caractère contre-productif et possiblement contraire au droit international du recours à ces armes, indiquant que les forces de l'ordre françaises comptent parmi les plus armées d'Europe. Bien évidemment, le recours à ces armes génère davantage de tensions et troubles à l'ordre public qu'il n'y apporte de solution. À moyen et long termes, le recours à des armes de plus en plus offensives participe de l'accroissement du niveau de violence et concourt à creuser le fossé entre les forces de sécurité et la population », estime estime l'ACAT. Une question s'impose : ces armes sont-elles vraiment adaptées au maintien de l'ordre lors de manifestations ? Sont-elles indispensables ? Peut-être y aurait-il lieu de légiférer sur le sujet prochainement avec la même ardeur qui vous amène aujourd'hui à défendre ce genre de dispositifs, mes chers collègues. La parole

qui sont utilisées lors des manifestations sont le plus souvent non pas des armes répertoriées, mais des armes par destination. Dans une manifestation, une batte de base-ball n'est pas un accessoire de sport,

plan le fait de détenir une arme et celui de détenir des fusées ou artifices, ou d'en faire usage, dans une manifestation sur la voie publique ou à proximité immédiate pour un quantum identique : trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. C'est inutile, car on vise tout objet susceptible de constituer une arme, alors que le port d'une par destination peut déjà être sanctionné. C'est redondant, car on propose de sanctionner le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité publique des personnes dans une manifestation sur la voie publique, alors que cet acte est poursuivi et réprimé par l'article 222-13 du code pénal en vigueur. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Cette modification ne paraît pas utile dans la mesure où le port, la détention ou l'introduction d'armes lors d'une manifestation peuvent déjà être réprimés par l'infraction actuelle de l'article 431-10 du code pénal, qui sanctionne largement le fait de participer à une manifestation en étant porteur d'une arme. De même, les précisions apportées quant aux objets pouvant servir d'armes- fusées ou artifices de toute nature -sont également inutiles, dès lors que l'article 132-75 du code pénal, auquel il est d'ailleurs fait renvoi, définit l'arme par destination comme tout objet dont l'utilisation ou la destination est susceptible de créer un danger pour les personnes.

Désormais, si l'article 5 est adopté, une personne détenant ou faisant usage de fusées ou artifices dans une manifestation sur la voie publique ou à proximité immédiate ou une personne porteuse d'une arme se trouvant dans les mêmes conditions seront toutes deux

Il est vrai que l'article 5 procède pour partie à une réécriture de l'article 431-10 du code pénal, qui explicite notamment la notion d'arme par destination. Il comporte cependant deux autres mesures plus substantielles auxquelles nous sommes attachés. D'une part, l'article 431-10 du code pénal sanctionne uniquement le port d'arme dans une manifestation. Nous proposons d'élargir un peu le champ de l'infraction en visant aussi les abords de la manifestation. En effet, les personnes à l'origine des débordements ne participent pas nécessairement à la manifestation, mais peuvent se trouver en marge part, la proposition de loi prévoit de sanctionner les tentatives de ces délits. Quelqu'un qui tenterait de jeter un projectile sur la foule ou sur les forces de l'ordre, mais qui s'en trouverait empêché, pourrait ainsi être poursuivi et sanctionné.

liées à l'organisation ou à la participation à une manifestation, et à renforcer la peine complémentaire d'interdiction de manifester. Encore une fois, plutôt que de durcir notre droit pénal et de porter atteinte aux libertés fondamentales, il serait temps de donner de vrais moyens à nos forces de l'ordre pour qu'elles exercent un travail de démantèlement en amont,

ont besoin de moyens supplémentaires pour assumer au mieux les missions de service public qui sont les leurs. Pour nous, la réponse au démantèlement de groupuscules tels que les Black Blocs ne réside sûrement pas dans l'accroissement des pouvoirs de police administrative ou dans le durcissement de notre droit pénal. Toutes les mesures de cette proposition de loi seront soit inefficaces, soit dangereuses pour nos libertés publiques. En outre, comme l'indique le rapport, l'interdiction de manifester n'est que très peu prononcée : entre 1995 et 2017, seules 32 condamnations ont été assorties d'une peine complémentaire d'interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique. Par ailleurs, aucune condamnation n'a été prononcée pour non-respect de cette interdiction. Aussi, au-delà de l'affichage politique, pourquoi s'acharner à durcir toutes les peines existantes

sur l'article. Si toute analogie avec les périodes sombres de l'histoire est particulièrement déplacée, on peut faire une analogie avec la façon dont nous parvenons à maîtriser et à réduire le phénomène du hooliganisme. Certes, les policiers demandent- nous les avons entendus ensemble, madame Assassi, au sein de la commission d'enquête parlementaire -plus de moyens matériels, humains, informatiques, mais ils demandent aussi plus de moyens juridiques. On entend On entend souvent dire qu'il faut renforcer et favoriser la prévention plutôt que la répression. La meilleure prévention en matière de dérapage dans les manifestations, c'est justement d'empêcher les casseurs répertoriés de s'y introduire

de manifester pour des casseurs déjà éprouvés est particulièrement bienvenue. J'entends parfois dire que cela n'a pas empêché le hooliganisme, mais je puis vous assurer, au nom de tous les élus confrontés à ce problème, que, si les dispositions législatives actuelles n'existaient pas et n'étaient pas mises en oeuvre, le phénomène de hooliganisme serait aujourd'hui bien plus important dans les stades. Certes, aucune disposition n'éteindra complètement un phénomène, mais ne pas mettre en oeuvre des dispositions nouvelles quand un phénomène comme celui-là est croissant nous interdit de le juguler. en oeuvre ce qui fonctionne contre le hooliganisme pour assurer un peu plus de sérénité dans les manifestations, au bénéfice premier des manifestants et au bénéfice second de tous nos concitoyens, notamment des riverains.

qui confirment l'orientation sécuritaire de ce texte. Nous ne sommes persuadés ni de leur efficacité ni de leur caractère opératoire. Je suis en désaccord complet avec ce qui vient d'être dit par M. Grosdidier sur le hooliganisme, j'ai eu l'occasion de l'évoquer lors de la discussion générale. Face à la

vous proposez d'alourdir des dispositifs qui ne les contrarieront en rien et qui ne le dissuaderont pas ! Par conséquent, l'extension du champ d'application de la peine complémentaire, la modification de la peine et l'application des peines complémentaires prévues pour le délit de port d'arme ne sont pas, à nos yeux, des améliorations de nature à éviter les phénomènes violents que vous pensez combattre.

puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, ou le nouveau délit créé par la proposition de loi de dissimulation de son visage dans une manifestation. Plus encore, cet article étend le champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de séjour à ces mêmes délits, ce qui est également disproportionné au regard des peines principales encourues. Au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1995, qui indique que l'équilibre à trouver par le législateur entre ordre public et garantie des libertés constitutionnellement protégées quand il crée une peine portant restriction de la liberté d'aller et venir est fonction non seulement de la fixation de lieux déterminés où la peine s'applique et du pouvoir du juge de décider de prononcer la peine ainsi que de son champ d'application, mais aussi de la nature des infractions pour lesquelles

L'extension du champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique mérite d'être tempérée par une exigence de proportionnalité, au risque d'entraver la liberté constitutionnelle d'aller et de venir. Vous venez de rappeler la décision du Conseil constitutionnel, monsieur le secrétaire d'État. Il nous incombe donc d'assurer la bonne articulation des exigences de l'ordre public et de la garantie des libertés constitutionnellement protégées.

des magistrats. La commission des lois considère l'extension des peines complémentaires proposée dans cet article comme un outil de prévention de la récidive de ces infractions. De plus, l'obligation de pointage renforce l'efficacité de ces peines. Cette disposition nous paraît particulièrement utile. Une telle extension n'est pas disproportionnée, parce qu'il s'agit de l'extension de la peine complémentaire de manifester ou de la peine d'interdiction de séjour.

L'article 6 est donc conforme en tout point à la décision du Conseil constitutionnel de 1995. Concernant la peine complémentaire d'interdiction de séjour, qui appelle une peine principale plus lourde, selon le Gouvernement, je rappelle, monsieur le secrétaire d'État, que cette peine est d'ores et déjà applicable à des délits punis d'une faible peine d'emprisonnement. Voici quelques exemples : cette peine complémentaire est applicable au délit de demande de fonds sous contrainte, qui est puni de six mois d'emprisonnement. Ce délit a été créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 mars 2003. La peine complémentaire d'interdiction de séjour est également applicable pour le délit prévu à l'article 431-22 du code pénal, pénal, lequel réprime d'une peine d'un an d'emprisonnement le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans autorisation. scolaire sans autorisation. Ce délit et les peines complémentaires afférentes créés par la loi du 2 mars 2010- je rappelle que cette loi renforce la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public -ont également été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans une décision du 25 février 2010. En conséquence, mes chers collègues, l'application de cette peine complémentaire à des infractions punies d'un an d'emprisonnement n'est pas disproportionnée et apparaît conforme

avec une tradition du Gouvernement, celle de rejeter les propositions de loi extrêmement pertinentes du Sénat. Le Gouvernement s'étant engagé à moins de verticalité,

que certains vivent dans ce merveilleux pays qu'est la théorie, où l'on intellectualise le monde, où l'on ne voit pas la réalité, où l'on ne perçoit pas que la démocratie peut parfois être fragilisée. Il m'est arrivé pendant les graves manifestations contre la loi Travail de me trouver à Rennes. Il est dommage que nous n'ayons pas été plus nombreux à arpenter cette ville le samedi matin.

que notre démocratie, qui est aujourd'hui très fragilisée, ne doit pas faire preuve de faiblesse. Elle doit protéger la liberté individuelle, mais aussi s'affirmer. Je salue donc le travail de protection des libertés individuelles

et nous sommes pour l'ordre républicain. La parole est à M. Bruno Retailleau,

une réponse à un phénomène qui devient extrêmement préoccupant. Je remercie donc le président de la commission des lois et la rapporteur d'avoir ajusté les dispositifs

du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites

il y a quasiment un an jour pour jour, j'étais devant vous pour l'examen de ce texte en tant que ministre auprès du ministre de l'intérieur. Aujourd'hui, c'est au titre de mes nouvelles responsabilités ministérielles que je me présente devant vous à l'occasion de la deuxième lecture de cette proposition de loi, dont le Sénat a souhaité la discussion. Certes, cette révision du cadre juridique applicable aux conditions d'accueil et d'habitat des gens du voyage- cadre issu de la loi du 5 juillet 2000 -aurait pu demeurer du ressort du ministère de l'intérieur. Il nous a toutefois semblé qu'elle s'inscrivait pleinement dans la démarche que je souhaite poursuivre, dans le cadre de ce ministère aux compétences élargies, qui est de placer les territoires et les collectivités qui les administrent au coeur de nos préoccupations. Cette proposition de loi répond parfaitement à cette volonté. Il m'a donc semblé naturel, dans le cadre de mes nouvelles fonctions, de poursuivre- d'achever, je l'espère -ce travail avec vous, dans un esprit constructif, comme je m'y étais engagée l'année dernière. J'en viens maintenant au fond du sujet. Cette proposition de loi répond à un besoin qui remonte des territoires. La Haute-Savoie est particulièrement touchée par cette situation, ce qui explique que M. Loïc Hervé et, à l'époque, M. Jean-Claude Carle nous aient proposé les dispositifs que nous étudions aujourd'hui.

j'entends l'exaspération qui en résulte et la volonté de légiférer pour mieux lutter contre certaines pratiques inacceptables. Je tiens tout d'abord à souligner que l'installation de la grande majorité de familles de gens du voyage se fait sans problème, sur des aires prévues à cet effet. En revanche, pour une minorité de cas, qui choisit l'installation illicite, la situation est problématique et peut conduire à des débordements, voire à des violences. C'est pourquoi nous avons demandé aux préfets d'utiliser pleinement les outils juridiques dont ils disposaient afin de mettre un terme à ces situations quand elles se présentaient. Ces installations illicites ont ainsi lieu sur tout type de terrain, agricole ou municipal, ou dans des zones industrielles. Elles empêchent l'utilisation du bien et pénalisent l'activité économique, créent des troubles et suscitent un profond mécontentement et des tensions avec les les propriétaires, la population et les élus. Il convient aussi de rappeler, et je sais que vous y êtes sensibles, que les gens du voyage doivent être accueillis dans de bonnes conditions, conformément à ce qui est prévu dans le cadre des prescriptions des schémas départementaux, et sur des aires d'installations géographiques adaptées à leurs besoins. Actuellement, dix-neuf départements sont à ce titre en parfaite conformité avec les obligations découlant des schémas. C'est une bonne chose, mais c'est encore insuffisant à l'échelon national, le taux de réalisation du total des prescriptions des schémas départementaux

ou à celles dans lesquelles il n'y a pas d'acceptation par les riverains de l'installation d'une aire près de chez eux. Toutefois, c'est grâce à un accueil adapté aux besoins des gens du voyage et à ce qui les caractérise- leur liberté de déplacement -que nous réunirons les conditions permettant de limiter les installations illicites, d'une minorité qui, on le sait, ne rentre jamais dans le cadre. Le respect du mode de vie des gens du voyage est un impératif, au même titre que la qualité de vie des personnes qui se trouvent aujourd'hui confrontées à ces installations. C'est à nous, collectivement, de donner à chacun les moyens de vivre sereinement la vie ou l'activité qu'il a choisie. Cela étant rappelé, le texte qui nous occupe aujourd'hui a pour objectif de renforcer et de corriger la loi au regard des cas particuliers qui tendent malgré tout à se multiplier. Lors de la première lecture, nous n'étions pas parvenus à un accord, et il était apparu un écart sensible entre ce que vous souhaitiez et ce que le Gouvernement était prêt à accepter. Je garde à cet égard un souvenir contrasté de la séance publique, puisque, malgré une approche plus que constructive de la part du Gouvernement, la Haute Assemblée n'avait souhaité écouter aucune des observations que j'avais alors formulées, votant ainsi le texte dans une version maximaliste, contenant des dispositifs que le Gouvernement avait jugé inopportuns ou peu opérationnels. Le groupe LR de l'Assemblée nationale ayant décidé d'inscrire à son ordre du jour réservé la discussion de cette proposition de loi adoptée par le Sénat, c'est dans le même état d'esprit que le Gouvernement en a abordé l'examen. J'ai ainsi plaidé auprès des groupes de la majorité parlementaire, qui m'ont entendue, afin qu'ils fassent preuve de la même approche constructive et approuvent des dispositifs qui allaient dans le sens d'un meilleur respect des obligations par les communes et d'une plus grande efficacité des procédures de lutte contre les installations illicites. Même si les députés ont dû s'y reprendre à deux fois pour des motifs sur lesquels je n'épiloguerai pas- les élus de Haute-Savoie savent ce qu'il en est -, l'Assemblée nationale a adopté cette proposition de loi le 21 juin dernier, dans des termes qui recueillent l'accord du Gouvernement. Même si je peux comprendre que d'aucuns regrettent la disparition de certains dispositifs avec lesquels le Gouvernement était en désaccord, je souscris néanmoins à la position de votre commission des lois. Sous l'impulsion de son rapporteur, Catherine Di Folco, dont je tiens à saluer le travail de grande qualité

Ce texte me paraît en effet représenter un compromis satisfaisant. La clarification des compétences des communes et de leurs groupements en matière d'accueil des gens du voyage, établies par la loi du 5 juillet 2000, était nécessaire, vous avez raison. En effet, les transferts de compétences nés de la loi MAPTAM et de la loi NOTRe ne s'étaient pas accompagnés des aménagements indispensables dans la loi Besson. Les EPCI étant désormais compétents en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires et terrains destinés aux gens du voyage, il s'avère que les obligations découlant des schémas départementaux reposent encore sur les communes, lesquelles, en vertu du principe d'exclusivité des compétences transférées, n'ont plus les outils pour agir. La proposition de loi, telle que présentée aujourd'hui, apporte donc cette clarification en matière de compétences pour chaque type de collectivités. J'entends également le besoin des communes d'accéder au pouvoir de police spéciale lorsqu'elles respectent leurs obligations, alors que ce pouvoir est aujourd'hui conditionné par le fait que l'EPCI remplisse l'intégralité des obligations qui lui incombent en application du schéma départemental. Leur incompréhension est légitime, et nous l'avons entendue. C'est pourquoi, afin de mieux lutter contre les installations illicites et de répondre aux besoins des élus qui, eux, ont mis en place des conditions d'accueil satisfaisantes sur le territoire de leur commune et se trouvent aujourd'hui

du 18 mars 2003 en cas d'occupation en réunion sans titre d'un terrain en vue d'y installer son habitation ainsi que l'application de la procédure de l'amende délictuelle forfaitaire sont des mesures qui me semblent aller dans le bon sens et être de nature à lutter efficacement contre les installations illicites. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement est à votre écoute et à celle des élus de vos territoires. Aucun sujet n'est pris à la légère, et mon implication sera totale quand vous me solliciterez, comme j'ai pu

à l'instar de votre commission des lois, à adopter ce texte sans modification. Très bien

Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, en première lecture par le Sénat le 31 octobre 2017, est issue de la fusion d'une proposition de loi de notre ancien collègue Jean-Claude Carle et d'une autre déposée par notre collègue Loïc Hervé. Elle avait pour objet d'apporter des réponses concrètes aux difficultés récurrentes provoquées, sur de nombreuses parties du territoire français, par l'occupation illicite de terrains publics ou privés. Il est en effet de la responsabilité de la puissance publique de garantir l'ordre public et les libertés des autres citoyens, en aménageant un juste équilibre des droits et des devoirs de chacun et en faisant cesser les agissements d'une minorité de fauteurs de troubles. L'Assemblée nationale a examiné le texte en juin et, malgré le rapport favorable fait au nom de la commission des lois par notre collègue députée Virginie Duby-Muller, que je remercie, nombre de dispositions pragmatiques et mesurées ont été purement et simplement supprimées, sans recherche de compromis. Ces dispositions utiles avaient plusieurs objets. Il s'agissait, d'abord, de mieux circonscrire les obligations susceptibles d'être assignées aux communes et à leurs groupements en matière d'accueil des gens du voyage, en prévoyant que le schéma départemental élaboré ne puisse imposer la réalisation d'aires ou de terrains d'accueil sur le territoire de communautés de communes ne comportant aucune commune de plus de 5 000 habitants. Il s'agissait, ensuite, de ne pas imposer la construction de nouvelles aires d'accueil ou de nouveaux terrains familiaux si les aires et terrains existants n'atteignaient pas un taux d'occupation minimal fixé par décret, ce qui nous semblait être juste du bon sens. Il s'agissait, encore, de comptabiliser en logements sociaux les emplacements en aire permanente d'accueil, à l'instar des terrains familiaux locatifs. Cela nous paraissait totalement justifié, compte tenu de la situation de précarité des personnes qui les occupent et des coûts importants d'aménagement et d'entretien incombant aux communes et à leurs groupements. Il s'agissait, en outre, de supprimer la procédure de consignation de fonds à l'égard des communes et EPCI défaillants, inutilement attentatoire à leur libre administration. Plutôt que d'imposer pareille procédure aux élus, l'État, à mon sens, ferait mieux de prendre sa juste part à l'amélioration des conditions d'accueil des gens du voyage. Je rappelle que, depuis 2009, il ne finance plus la réalisation des aires d'accueil et terrains familiaux, sauf pour les communes nouvellement inscrites au schéma départemental. Le montant de ses subventions est passé de 46 millions d'euros en 2008 à 5,3 millions d'euros en 2018. Le texte prévoyait également de relever le montant de la taxe sur les résidences mobiles occupées à titre d'habitat principal, afin de fournir un surcroît de recettes aux communes et EPCI qui construisent ces aires et ces terrains d'accueil.

la durée d'applicabilité de cette mise en demeure d'évacuer et de l'étendre à l'ensemble du territoire communal ou intercommunal, afin d'éviter la reconstruction immédiate de campements illicites à proximité. Sur ce sujet, l'opposition sans nuance de la majorité gouvernementale est désolante. Les procédures actuelles ont montré leurs limites, au point que des heurts violents éclatent, chaque année, entre les habitants, les agriculteurs ou autres entrepreneurs et les occupants illicites. N'est-il pas de la responsabilité du législateur d'aménager des voies de droit pour éviter que la voie de fait ne prenne le dessus ? Les mesures adoptées par le Sénat n'avaient rien d'excessif et auraient fourni des éléments de réponse aux attentes légitimes des élus et des citoyens. par ailleurs, prévu de renforcer la répression pénale des installations en réunion et sans titre sur un terrain, ainsi que des destructions et dégradations commises aux mêmes occasions, tout en veillant à ce que les mesures soient adaptées et proportionnées, dans le respect de la jurisprudence constitutionnelle. Ainsi, l'article 8 créait un délit d'occupation habituelle en réunion d'un terrain sans titre et l'article 9 instituait deux nouvelles peines complémentaires : l'interdiction de séjour et la confiscation des véhicules destinés à l'habitation. Toutefois, plusieurs dispositions importantes et urgentes ont été maintenues, parmi lesquelles figure une clarification de la répartition des compétences entre les communes et leurs groupements à fiscalité propre, rendue nécessaire par les dernières réformes territoriales. l'obligation d'information préalable des autorités publiques lors des grands passages et grands rassemblements de gens du voyage, ainsi que la possibilité, pour un maire qui ne serait pas en mesure d'assurer l'ordre public par ses propres moyens lors de ces grands rassemblements, de demander au préfet de département de prendre les mesures nécessaires. mesure très importante et attendue, vous l'avez rappelé, madame la ministre, à savoir l'extension au maire de toute commune dotée d'une aire ou de terrains d'accueil du pouvoir d'interdire le stationnement des résidences mobiles sur le reste du territoire communal. sera par conséquent possible de demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure d'évacuation d'office des campements illicites, même dans le cas où l'EPCI auquel la commune appartient n'a pas rempli l'ensemble de ses obligations. Cette mesure mettra fin à une interprétation aberrante de la loi et répondra à une attente ancienne des élus. Autre mesure conservée : le doublement des peines encourues en cas d'installation en réunion et sans titre sur le terrain d'autrui, et l'application à ce délit de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle, qui en facilitera la répression. Cette proposition de loi du Sénat nous revient donc en deuxième lecture, c'est assez rare pour être relevé, et nous avons abordé cette nouvelle étape avec un esprit partagé. Si un grand nombre de dispositions adoptées par le Sénat ont été supprimées, un début de solution est tout de même apporté au problème de stationnement illicite des gens du voyage. Nous ne sommes pas satisfaits ; il ne s'agit pas d'un compromis. Il faut aller plus loin pour répondre aux préoccupations légitimes des élus, sans doute à l'occasion d'un nouveau vecteur législatif. Pour l'heure, il me semble important de ne pas laisser passer l'opportunité de voir les mesures qui subsistent, toutes dues à l'initiative du Sénat, entrer en vigueur sans délai.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, l'heure semble venue de mettre fin au casse-tête et aux difficultés permanentes que constitue, pour les élus locaux, l'accueil des gens du voyage.

réglaient ces conditions d'accueil : la loi Besson, la loi MAPTAM, la loi NOTRe et la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Au fil de la navette, les règles et les responsabilités de chacun, notamment des communes et des intercommunalités, se sont précisées, sauf, et c'est plus que fâcheux, s'agissant des communes de moins de 5 000 habitants, que la loi Besson excluait de l'obligation d'accueil. D'où l'amendement de mon groupe, par lequel nous ne faisons d'ailleurs que reprendre une disposition adoptée par le Sénat en première lecture avant d'être supprimée, on ne sait pourquoi, par l'Assemblée nationale. Ne pas le voter serait accepter que des EPCI composés de petites communes, qui, jusqu'à ce jour, n'avaient pas d'obligation d'accueil, y soient directement soumis. Je constate que, décidément, l'esprit de la loi NOTRe souffle encore ... Plus encore qu'à l'enchevêtrement réglementaire, les difficultés actuelles tiennent à deux choses. Elles tiennent, premièrement, aux retards dans l'élaboration et la mise en oeuvre des schémas départementaux. si nous avions beaucoup avancé, 35 % des aires d'accueil permanentes restaient encore à réaliser. Surtout, 18 % de celles qui existaient alors ne répondaient pas complètement aux obligations prévues. J'espère que, depuis cette date, des progrès substantiels ont été faits.

à la perspective de faire évacuer par la force publique les contrevenants qui s'installent là où bon leur semble, parfois même quand existe une aire d'accueil réglementaire sur le territoire de la commune Si le présent texte précise les obligations et pouvoirs de chacun, ceux des maires notamment, il ne peut garantir une meilleure application desdites règles, application qui relève de l'ordre public et, donc, du pouvoir d'appréciation du préfet, en fonction des moyens des moyens dont il dispose, lesquels, vous le savez comme moi, ne sont pas toujours suffisants. En tout cas, ces retards, voire ces absences de réaction de la part des pouvoirs publics, sont source d'incompréhension pour les élus, de rejet par le voisinage, qui en vient à se demander s'il n'y a pas deux catégories de citoyens : ceux que l'on sanctionne quand ils ne respectent pas la loi et ceux qui peuvent tout se permettre en toute impunité. Voilà une particularité qui, d'ailleurs, je le souligne, n'est pas une exclusivité propre aux gens du voyage ; mais passons Notre sentiment est que nous ne sortirons de l'impasse qu'en faisant respecter la loi Besson et rien que la loi Besson, par les uns comme par les autres par les collectivités, en facilitant la réalisation des aires d'accueil ; par les gens du voyage, en facilitant la police des grands rassemblements ainsi que l'évacuation des terrains occupés illégalement dans les EPCI qui, eux, respectent la loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous débattons de nouveau au sein de notre hémicycle de la proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et et à la lutte contre les installations illicites, sensiblement modifiée par l'Assemblée nationale. Lors de son examen en octobre 2017, j'avais d'emblée regretté, au nom de mon groupe politique, que nous ayons à examiner un ensemble de mesures remettant en cause le dispositif équilibré et concerté voté au sein de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, dite loi LEC. Rappelons que cette loi a permis d'adapter et d'améliorer la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dite loi Besson, en précisant les conditions d'élaboration des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage et en renforçant les dispositifs de mise en demeure et d'évacuation des campements sauvages. Elle a en outre facilité le recours à la procédure du référé, afin de mieux protéger les terrains, notamment les terrains agricoles, lorsque l'activité économique est entravée. Dans le même temps, la LEC a abrogé des dispositions discriminantes, comme le livret de circulation et l'obligation qui était faite de le faire viser à intervalles réguliers par l'autorité administrative, ce dont je me félicite de nouveau. Elle a également réaffirmé le droit à la scolarisation des enfants du voyage et introduit une procédure de consignation de fonds à l'encontre des communes et EPCI ne remplissant pas les obligations du schéma départemental. Je veux le souligner de nouveau ici : en matière d'accueil des gens du voyage, l'enjeu aurait d'abord été d'appliquer la LEC et l'ensemble de la législation existante au lieu de proposer, comme c'était le cas initialement dans cette proposition de loi, un nouvel arsenal de mesures répressives, et pour certaines inapplicables, au risque de nous placer dans une simple logique d'affichage. Fort heureusement, le texte tel que nous l'examinons aujourd'hui se trouve désormais délesté de ses mesures les plus sujettes à caution, à la suite de son examen par l'Assemblée nationale en avril puis au mois de juin dernier. Je me félicite, tout d'abord, que les mesures dérogatoires en matière d'obligations d'accueil que souhaitait instaurer la majorité sénatoriale aient été supprimées. Il en est ainsi du caractère facultatif de la création d'installations d'accueil pour une commune appartenant à une communauté de communes dont aucune d'entre elles ne dépasse 5 000 habitants. supprimées : la comptabilisation des aires permanentes d'accueil des gens du voyage au sein des logements sociaux pour l'appréciation du respect de la loi SRU, ainsi que le rétablissement de la procédure de consignation de fonds introduite par la loi Égalité et citoyenneté à l'encontre des communes et EPCI ne remplissant pas les obligations du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. La navette parlementaire a également permis de supprimer un certain nombre de dispositions inutilement répressives à l'encontre des gens du voyage : l'augmentation de la taxe sur les résidences mobiles terrestres, ainsi que la création d'une vignette délivrée délivrée lors du paiement de la taxe avec obligation de l'apposer de manière visible sur le véhicule redevable ; l'instauration d'une peine complémentaire d'interdiction de séjour ajoutée à la peine principale qui serait prononcée au titre d'une occupation illégale de terrain ; la de terrain ; la possibilité de saisir des véhicules destinés à l'habitation. Dans le même temps ont été maintenues, au sein du texte, des mesures visant à répondre efficacement aux difficultés rencontrées par les collectivités territoriales. Pour le stationnement d'un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles, les représentants des gens du voyage devront dorénavant obligatoirement informer au moins trois mois avant le préfet de région, le préfet de département et le président de conseil départemental concernés. Le préfet de département avertira ensuite les élus locaux. Si le maire n'est pas en mesure d'assurer l'ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, il pourra demander au représentant de l'État dans le département de prendre les mesures nécessaires. En outre, une commune qui respecte ses obligations en matière d'accueil pourra interdire le stationnement en dehors des aires aménagées, même si elle appartient à un EPCI ne respectant pas, sur son territoire, les obligations qui lui sont faites dans le cadre du schéma départemental. les sanctions pénales en cas d'occupation en réunion sans titre d'un terrain sont renforcées, avec un doublement de la peine encourue, portée à douze mois d'emprisonnement et à 7 500 euros d'amende. Si cette dernière mesure nous laisse quelque peu dubitatifs, nous saluons en revanche l'instauration d'une amende forfaitaire délictuelle, d'un montant de 500 euros, qui stoppera l'action publique engagée tout en permettant la sanction immédiate de l'infraction commise. Je me félicite également que les compétences entre les communes et les EPCI aient été clarifiées et l'intercommunalité réaffirmée comme l'échelon pertinent en matière d'accueil des gens du voyage. La loi indiquera dorénavant que les communes sont tenues d'accueillir une installation, mais ce seront bien les EPCI qui devront assurer la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires et terrains prévus par le schéma départemental. Au vu de l'ensemble de ces modifications, je considère, au nom de mon groupe, que cette proposition de loi ainsi rédigée correspond davantage à l'approche équilibrée en droits et en devoirs que nous appelions de nos voeux et que nous avions d'emblée cherché à établir en déposant un certain nombre d'amendements en première lecture. En effet, nous sommes tout autant que vous, chers collègues de la majorité sénatoriale, conscients des difficultés auxquelles peuvent être confrontés les élus locaux en matière d'accueil des gens du voyage. Je tiens d'ailleurs de nouveau à leur rendre hommage dans cet hémicycle et à saluer leur action essentielle au service de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire. L'action et l'engagement des élus locaux sont précieux et indispensables au bon fonctionnement de notre République décentralisée. Nous devons donc leur donner les moyens d'agir, en leur fournissant, dans le cas présent, les outils législatifs adéquats pour pouvoir non seulement accueillir toutes les populations dans de bonnes conditions, mais également remédier aux situations d'occupations illicites et réprimer l'ensemble des comportements contraires à la loi. De même, nous savons qu'il est nécessaire que l'ensemble des collectivités se conforment à leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage.

et, à ce jour, seuls dix-huit départements respectent leurs obligations d'accueil. Nous devons tout faire pour améliorer ces chiffres et cette réalité statistique, qui ne peut nous satisfaire et doit nous interpeller. Pour les collectivités satisfaisant à ces obligations, il est essentiel que les terrains mis à disposition respectent les critères d'accueil élémentaire requis, tels que l'accès à l'électricité, à l'eau potable et à des conditions de vie décentes. Comme je l'ai rappelé lors de l'examen de ce texte en commission des lois, la question de l'accueil des gens du voyage ne se réglera pas par la seule inflation des sanctions. Adoptons une approche plus équilibrée, en nous souciant, par exemple, de l'accueil des enfants des gens du voyage dans les écoles, ou en prenant en considération les effets positifs que de tels rassemblements peuvent apporter en termes de brassage social ou de gain d'activité économique sur le territoire, notamment autour des aires de grand passage. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, nous ne sommes ici ni dans l'angélisme ni dans le tout-répressif. Nous souhaitons avant tout défendre un principe simple : le respect des droits et des devoirs de chacun. en somme, de faire confiance aux élus locaux, en leur donnant les moyens juridiques d'agir si nécessaire tout en défendant un accueil digne des gens du voyage, conforme à nos valeurs. De manière pragmatique et au vu des améliorations notables apportées au cours de la navette parlementaire, notre groupe politique votera donc en faveur de cette proposition de loi. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, le texte de loi examiné aujourd'hui, issu des propositions de loi déposées par notre ancien collègue sénateur Jean-Claude Carle et par notre collègue Loïc Hervé, entend répondre à une problématique sensible, rencontrée sur le terrain par nombre de nos élus locaux, qui se sentent impuissants, voire abandonnés par les services de l'État. la question du rôle des collectivités territoriales dans l'accueil des gens du voyage, dont le Sénat s'est saisi, revient à rechercher de façon constante un juste équilibre : un juste équilibre entre la liberté de mouvement de personnes itinérantes et le droit de propriété un juste équilibre entre les besoins spécifiques des gens du voyage et le maintien de l'ordre public ; un juste équilibre, aussi, dans la répartition des compétences entre les différentes collectivités territoriales et l'État. L'arsenal législatif en vigueur, constitué par la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dite loi Besson, et par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, a permis de poser le socle des droits et des devoirs qui incombent à chacun. qui concerne les collectivités locales, ces dernières ont l'obligation de mettre en place des aires d'accueil réservées pour les itinérants, afin de favoriser leur intégration. les gens du voyage sont tenus de respecter les règles collectives, en vue de prévenir la dégradation de lieux publics et l'occupation illégale de terrains. Mais certains dispositifs se sont révélés trop complexes, voire inadaptés aux réalités du terrain, face notamment au phénomène de semi-sédentarisation ou de sédentarisation des gens du voyage. Il était donc devenu urgent d'apporter des solutions concrètes, à la hauteur des attentes de nos élus, qui sont fortes. C'est pourquoi le groupe du RDSE soutient les dispositions contenues dans ce texte, dotant les maires de nouveaux outils juridiques pour faire respecter le droit commun et l'ordre public.

Cette mesure très concrète est cruciale pour les élus. Elle leur permet de s'organiser pour faire face à des afflux importants de population et de véhicules, ce qui est le minimum quand on sait que, lors de ces grands rassemblements, ce sont des centaines de personnes, voire des milliers, qui peuvent se réunir sur un même lieu pour une quinzaine de jours. Je citerai en exemple une situation que je connais bien, ayant lieu tous les ans dans mon département girondin : un grand rassemblement de gens du voyage à caractère religieux y regroupe 3 000 itinérants sur le territoire d'une commune de 2 400 habitants. Un tel mouvement de personnes implique un certain nombre de bouleversements, qu'il convient, comme vous pouvez l'imaginer, d'anticiper. En termes sanitaires, il s'agit notamment de prévoir l'évacuation des déchets et l'alimentation en eau. Je pense aussi aux milieux sensibles, qu'il faut protéger, à l'instar de la forêt des Landes girondines. Il est indispensable de protéger notre réseau de pistes DFCI- défense des forêts contre l'incendie -, dont les règles de circulation sont respectées au quotidien par la population résidente. Il faut donc nous assurer

quand un grand rassemblement a lieu lors de la période cruciale de l'ouverture de la chasse, des réunions préparatoires sont absolument indispensables entre les services locaux et ceux de l'État, et ce suffisamment en amont. le texte prévoit la possibilité pour les maires de demander au préfet de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, quand ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de le faire. Cette proposition de loi permet aussi aux communes dotées d'une aire d'accueil de prendre des arrêtés d'interdiction de stationnement, afin que les maires ne soient plus pénalisés par les manquements des EPCI, dont leur commune est membre.

l'article 1 répond à une forte attente de clarification des compétences entre les communes et les EPCI et permet de mieux prendre en compte les nouvelles compétences des intercommunalités. Si ce texte renforce la responsabilité des collectivités locales en termes d'accueil des gens du voyage, il permet de leur assurer aussi qu'elles ne sont pas seules. L'État doit être garant de cet équilibre et acteur d'une solidarité territoriale. Le chantier est de taille

que 25 % d'entre elles n'utilisent pas les outils de suivi de scolarité, dispositifs pourtant clés dans le cas d'une scolarité en itinérance. Si les obligations des collectivités doivent être évidemment respectées, l'État ne peut se détourner des siennes. Concernant le renforcement des sanctions contre les occupations illicites, sujet sur lequel a particulièrement travaillé notre collègue Loïc Hervé, certains membres du groupe du RDSE émettent des réserves techniques quant au doublement des sanctions pour l'occupation d'un terrain sans titre ou la création d'une amende forfaitaire délictuelle en cas d'occupation illicite. Ces interrogations techniques reposent sur le fait que la justice et la police, confrontées à des tâches nombreuses et fournies, pourraient dans les faits ne pas se saisir de ces outils. En tout état de cause, cette disposition est maintenant introduite dans le texte, et nous pouvons compter sur la ténacité des élus pour la faire appliquer. En conclusion, le groupe du RDSE tient à saluer le compromis trouvé entre les deux chambres du Parlement dans l'examen de ce texte, qui soulève des problématiques éminemment complexes et clivantes. Au fil des lectures, le Sénat et l'Assemblée nationale ont travaillé à la poursuite d'un juste équilibre, fortement attendu par les élus locaux. Néanmoins, pour aboutir à ce compromis, il a fallu faire des concessions : il est regrettable que l'article 2 prévoyant l'abrogation de la procédure de consignation de fonds à l'égard des communes et des EPCI défaillants ait été supprimé à l'Assemblée nationale. Lors de la première lecture, les membres du RDSE avaient conditionné leur vote final à l'adoption des amendements déposés par le groupe.

un an après le vote d'un texte au Sénat, nous sommes amenés à débattre à nouveau ce soir, en deuxième lecture, de la question de l'accueil des gens du voyage et de la lutte contre les installations illicites. Comme auteur de l'une des deux propositions de loi initiales, tout comme l'était notre ancien collègue Jean-Claude Carle- Cyril Pellevat en était le premier signataire -, je me sens une responsabilité particulière dans ce débat. En effet, chacun ici a conscience que la situation reste critique, et l'année qui s'est écoulée n'a pas vu d'amélioration. Les entreprises, les agriculteurs, les élus locaux, les forces de l'ordre, les magistrats sont, pour nombre d'entre eux, épuisés et et exaspérés par des situations qui durent et se répètent. Il faut entendre cet appel à l'aide et y répondre autant que possible. À titre d'exemple, je pourrais vous parler de la Haute-Savoie, où les maires réunis en congrès départemental samedi dernier ont encore manifesté leur ras-le-bol, publiquement et ouvertement.

si les auteurs des propositions de loi sont haut-savoyards et les sénateurs de ce département particulièrement vigilants sur ce sujet, la question se pose dans tout le pays. En témoignent les très nombreux collègues cosignataires de nos propositions

aussi depuis lors. C'est grâce à vous, chère collègue, que le Sénat a adopté un texte cohérent et robuste que l'Assemblée nationale, lors de son examen, a malheureusement soulagé de nombreuses propositions importantes. Si l'on peut émettre des regrets, je voudrais à cet instant souligner, madame la ministre, que votre oreille a toujours été attentive et votre rôle positif, à la fois quand nous vous avons rencontrée place Beauvau, quand vous êtes venue dans notre département, en particulier dans le Genevois, et quand nous avons été amenés à évoquer ensemble ce texte et son destin. Alors, mes chers collègues, je voudrais vous faire part de mon état d'esprit ce soir. Je voudrais d'abord regretter les mesures que nos collègues députés n'ont pas conservées.

J'ai entendu, madame la ministre, que vous compreniez ce besoin, et c'est quelque chose que nous pourrons entreprendre au Sénat avec les collègues qui le souhaiteront. Il y a aussi les mesures conservées.

Mes chers collègues, à quelques jours du congrès des maires, notre vote permettra d'envoyer un signal clair aux élus de tout le pays : le Sénat s'est de nouveau

ce texte, issu de deux propositions de loi déposées respectivement par notre ancien collègue Jean-Claude Carle et notre collègue Loïc Hervé, a pour objet d'apporter des réponses concrètes aux difficultés récurrentes

à simplifier la préparation des grands passages et des grands rassemblements, à renforcer les moyens dont disposent les autorités publiques pour réglementer le stationnement des résidences mobiles, à faciliter l'évacuation des campements irréguliers et à mieux réprimer certains comportements. Il n'est pas question ici de jeter un quelconque discrédit ou de stigmatiser une catégorie de la population, mais il est de la responsabilité de la puissance publique de garantir l'ordre et les libertés des citoyens sédentaires, en aménageant un juste équilibre entre les droits et devoirs de chacun et en faisant cesser les agissements d'une minorité de fauteurs de troubles.

Je regrette ainsi la suppression d'un grand nombre de dispositions, pourtant utiles, proposées par le Sénat, notamment celle qui visait à supprimer la procédure de consignation de fonds à l'égard des communes et des EPCI défaillants, inutilement attentatoire à leur libre administration. Je désapprouve également la suppression par l'Assemblée nationale des dispositions qui avaient pour objet de mieux circonscrire les obligations susceptibles d'être assignées aux communes et à leurs groupements en matière d'accueil des gens du voyage, en prévoyant que le schéma départemental élaboré à cet effet ne puisse imposer la réalisation d'aires ou de terrains d'accueil sur le territoire de communautés de communes ne comportant aucune commune de plus de 5 000 habitants ou en cas de faible occupation des aires existantes. Je regrette aussi que l'Assemblée nationale ait amputé ce texte de mesures pertinentes. J'en citerai trois : le relèvement du montant de la taxe sur les résidences mobiles occupées à titre d'habitat principal la simplification de l'évacuation des campements illicites grâce au renforcement des procédures administratives et juridictionnelles ; enfin, le renforcement de la répression pénale des installations en réunion et sans titre sur un terrain, ainsi que des destructions et dégradations commises aux mêmes occasions, en instituant notamment une nouvelle peine complémentaire de confiscation des véhicules destinés à l'habitation. Toutefois, plusieurs dispositions importantes et urgentes ont été maintenues, et je m'en réjouis. Je citerai notamment la clarification de la répartition des compétences entre les communes et leurs groupements à fiscalité propre et l'obligation l'obligation d'information préalable des autorités publiques lors des grands passages et grands rassemblements de gens du voyage. Il faut aussi noter l'extension au maire de toute commune dotée d'une d'une aire ou de terrains d'accueil du pouvoir d'interdire le stationnement des résidences mobiles sur le reste du territoire communal et, par conséquent, de demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure d'évacuation d'office des campements illicites, même dans le cas où l'EPCI auquel la commune appartient n'a pas rempli l'ensemble de ses obligations. Je citerai enfin le doublement des peines encourues en cas d'installation en réunion et sans titre sur le terrain d'autrui et l'application à ce délit de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle, qui en facilitera la répression.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues- cher Loïc Hervé -, une proposition de loi du Sénat nous revient en deuxième lecture. Je n'ai pas une grande expérience de cet hémicycle, mais je crois que c'est suffisamment rare pour le souligner. Il faut aussi souligner la sagesse de Mme la rapporteur,

je suis d'accord avec d'autres. S'agissant de l'article 1, j'avais exprimé ma circonspection quant à exclure du schéma départemental près de la moitié des intercommunalités, celles qui ne comptent aucune commune de plus de 5 000 habitants.

nous pouvons nous réjouir de la clarification, nécessaire, de la répartition des compétences entre communes et EPCI, qui inclut la création des aires et terrains d'accueil dans les obligations des EPCI. Je partage le regret de ne pas avoir pu maintenir la suppression de la procédure de consignation de fonds à l'encontre des EPCI défaillants, procédure qui, en effet, pose la question de l'application du principe de libre administration des collectivités territoriales. L'article 3 est une avancée pour les élus locaux, qui pourront, grâce à ce mécanisme d'information préalable, s'organiser pour accueillir les gens du voyage lors des grands passages et des grands rassemblements. De même, l'article 4 satisfait aux préoccupations des élus, que le Gouvernement a entendues. Désormais, les maires d'une commune dotée d'une aire d'accueil pourront interdire le stationnement des résidences mobiles sur le reste du territoire communal, même si l'intercommunalité n'a pas satisfait à ses obligations.

La suppression par nos collègues députés de la confiscation des véhicules d'habitation me paraît conforme au principe d'inviolabilité du domicile. J'avais exprimé mes réserves sur cette disposition en première lecture. L'arsenal pénal existant pour réprimer les destructions, dégradations ou détériorations d'un bien d'autrui étant suffisant selon plusieurs avis recueillis, il ne nous paraissait pas indispensable de le renforcer. La suppression de l'article 7 par l'Assemblée donc nous convenir. L'article 8, qui prévoit la création d'un délit de fraude d'habitude d'installation, s'il n'est pas dépourvu de fondement,

Je vous souhaite de réussir pleinement votre mission pour le bien-être de nos collectivités, vous savez qu'elles attendent beaucoup ! Je suis heureux de voir- enfin -revenir au Sénat cette proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage, après un an d'attente. suis aussi très déçu de la réduction de son contenu. L'Assemblée nationale a supprimé les deux tiers des dispositions de notre texte. J'en déduis que l'ampleur de la situation sur le terrain est clairement sous-estimée par certains députés. Je l'ai maintes fois répété : en Haute-Savoie, comme dans bien d'autres départements, nous sommes assis sur une véritable poudrière, qui peut s'embraser à tout moment. Les exemples d'altercation avec les élus et les agriculteurs sont trop nombreux. Non, nous ne stigmatisons pas les gens du voyage, comme cela a pu être dit sur les bancs de l'Assemblée nationale ! Nous faisons une différence entre les gens du voyage qui respectent les règles- ils représentent une très large majorité -et ceux qui, au contraire, se comportent comme des délinquants et ne respectent ni les lois de la République ni les arrêtés des communes ou des EPCI. Bref, des vrais-faux gens du voyage, qui restent sur un périmètre d'une trentaine de kilomètres ! Ce sont ces derniers qui posent problème. Avec mes deux collègues sénateurs, Loïc Hervé et Sylviane Noël, nous nous faisons les porte-parole des nombreux élus qui subissent des installations illicites, sans disposer de réels moyens d'action, et qui nous interpellent régulièrement tout au long de l'année. Les installations n'ont pas seulement lieu pendant l'été ; elles se font durant des périodes qui sont de plus en plus longues, et la tension monte en puissance, allant parfois jusqu'à des incidents majeurs, comme nous en avons connus en Haute-Savoie où un maire et un gendarme Madame la ministre, les élus du territoire et les services de l'État sont investis dans leurs missions. La plupart des élus respectent les obligations légales décidées dans le cadre du schéma départemental des gens du voyage, mais certains groupes semblent s'affranchir des droits fondamentaux, tels que le droit de propriété, qui est régulièrement bafoué. Des groupes se sont imposés dans le département par le nombre et la force, bien qu'un refus de séjour leur ait été notifié en début d'année, puis réitéré lorsqu'ils se sont annoncés la veille pour le lendemain. D'autres arrivent aussi à leur convenance, méconnaissant les dates officielles de réservation. Les élus locaux sont condamnés à passer nuit et jour à gérer les installations illicites, à subir les invectives, les menaces, les intimidations et à constater des dégradations sur des terrains de foot ou des aménagements municipaux, sans jamais pouvoir se retourner contre ceux qui dégradent volontairement ces espaces. Ils doivent aussi gérer les interrogations de la population, qui fustige une justice à deux vitesses et estime nos lois trop permissives. Les propriétaires de terrains privés, chefs d'entreprise ou particuliers, ne comprennent pas que l'on puisse s'installer en toute impunité sur leur terrain et qu'il leur revient d'entamer des procédures longues et coûteuses. Les agriculteurs subissent des dégradations de leur outil de travail avec toutes les nuisances que cela entraîne : pertes de récoltes, dégâts dans les champs dus aux détritus- lames de rasoir, déchets plastiques, etc. -qui peuvent nuire aux appellations d'origine contrôlée Nous sentons également sur le terrain l'exaspération des forces de gendarmerie, qui sont mobilisées avec des effectifs limités, face à de grands groupes et pendant des périodes de plus en plus longues. Devant ce constat, tous les acteurs concernés espéraient un vote rapide et conforme dans chaque chambre. La proposition de loi n'était pas partisane et comportait des mesures utiles. Je souhaite remercier, à cet instant, ma collègue Catherine Di Folco pour la qualité de son rapport. Malheureusement, l'examen à l'Assemblée nationale fut surprenant : le texte a été entièrement détricoté. La proposition de loi qui nous revient en deuxième lecture est donc bien différente de celle que nous avions votée. Les députés de la majorité ont choisi de la vider en grande partie, je ne peux que le regretter. je soutiens pleinement les quelques dispositions qui restent, car elles constituent des avancées. J'insiste sur ce point : la situation est si critique que nous devons adopter ces mesures

Il est donc plus que nécessaire d'adopter ce texte et de veiller à son application. Les quatre mesures qui constituent cette proposition de loi comblent un vide législatif et apportent des réponses concrètes. Je ne vais pas les détailler, mais soyez

Je regrette bien sûr que n'ait pas été retenue par les députés la possibilité que nous avions donnée aux communes de moins de 5 000 habitants de ne pas installer d'aires d'accueil, hormis si elles étaient membres d'un EPCI comportant au moins une commune dépassant ce seuil.

nous espérons davantage de compréhension. Nous devons avoir le courage de nous retrouver, tous partis confondus, lorsqu'il s'agit de soutenir les élus locaux. La parole est à M.

ce mode de vie doit s'exercer dans le respect des lois de la République. En séance publique, les députés de la majorité présidentielle ont affirmé que « les manquements persistants concernant la réalisation d'aires d'accueil ont pour conséquence une installation massive sur des emplacements illicites S'il y a des occupations illicites, c'est donc la faute des communes, qui n'auraient pas réalisé un nombre d'aires d'accueil suffisant. Le raccourci était facile, la situation est bien plus complexe Dans la métropole Tours Val de Loire, où je suis élu, le taux d'occupation des aires d'accueil était d'environ 47 % en 2017. La même année, un minimum de 150 caravanes était identifié sur le territoire de la métropole en stationnement illicite durable. N'est-il pas totalement ubuesque de continuer à imposer des investissements supplémentaires aux collectivités, alors que les aires existantes sont occupées à moins de la moitié de leurs capacités ? ajouter à cet investissement les sommes déboursées pour entretenir les aires existantes, engager les procédures judiciaires d'expulsion des occupations illicites, puis nettoyer et réhabiliter les lieux libérés. Serait-il totalement incohérent de corréler la réalisation des aires d'accueil au taux d'occupation de celles qui existent ? Rappelons qu'une partie de la subvention versée par l'État est elle-même calculée en fonction de ce même taux d'occupation. De plus, pourquoi une commune respecterait-elle ses obligations et poursuivrait-elle son effort si, malgré des investissements colossaux, les campements illicites perdurent et sont même en constante augmentation ? Plus encore, comment expliquer au contribuable qu'il vaut mieux investir dans une aire d'accueil inoccupée plutôt que dans un service public de proximité ? Comment lui expliquer que, s'il est mal garé, il paiera une amende et que sa voiture partira sur-le-champ à la fourrière, mais qu'il faudra plusieurs semaines pour faire cesser une occupation illicite de gens du voyage qui, finalement, s'installeront cent mètres plus loin ? La population est excédée ; le climat devient délétère. Dépourvus de moyens d'action, abandonnés par l'État, les maires font l'objet d'attaques verbales, parfois physiques. Cet été, dans mon département d'Indre-et-Loire, réputé paisible, comme le Loir-et-Cher, madame la ministre, à Luynes plus précisément, 200 caravanes ont occupé les terrains de sport. Le maire de cette commune, qui avait investi 800 000 euros dans une aire d'accueil, a été la cible de jets de pierre, de coups de poing et s'est fait bousculer par une voiture. Tel autre maire, à Neuillé-Pont-Pierre, a subi une hospitalisation de huit jours après avoir été molesté par des gens du voyage à qui il demandait d'évacuer un terrain communal. Ce climat contribue à alimenter l'amalgame que peut faire la population entre les auteurs de ces pratiques illicites, dangereuses, et la grande majorité des gens du voyage, dont l'installation sur les aires d'accueil n'engendre pas de troubles. Non seulement l'effort de construction de places d'accueil doit être corrélé au taux d'occupation des aires existantes, mais sa contrepartie doit être l'évacuation rapide des campements illicites.

permettre aux policiers, aux gendarmes, aux élus locaux de cesser d'être de simples spectateurs de ces occupations illicites, dépourvus de tout moyen d'action, et de redevenir acteurs. L'État de droit existe lorsque la loi votée par le Parlement est appliquée et que les décisions administratives sont rapidement exécutées. La majorité gouvernementale a cependant voulu que, sur les dix articles que comportait la proposition de loi sénatoriale, il n'en reste que quatre. Selon l'aveu de Mme la rapporteur de la commission des lois, seule une adoption conforme de ces quatre articles, minimalistes, mais essentiels, permettra de donner une réponse rapide aux élus locaux.

en dépit de la généralisation d'aires d'accueil des gens du voyage dans les communes depuis de nombreuses années, les installations illicites demeurent un problème récurrent, à l'origine de lourds dommages aux propriétés publiques et privées, ainsi que de tensions parfois vives entre riverains et gens du voyage. Tous ces efforts, tous ces investissements coûteux pour rien », nous disent nos collègues maires et élus. « À quoi bon, si la loi n'est pas respectée ? », ajoutent-ils. Voilà tout juste un an, la proposition de loi de mon prédécesseur, Jean-Claude Carle, était adoptée à une très large majorité par le Sénat. Inscrit dans une niche parlementaire du groupe Les Républicains, ce texte répondait en effet aux attentes fortes des élus locaux, régulièrement démunis face à certaines occupations illicites. Cette proposition de loi a malheureusement été vidée de sa substance en première lecture par le groupe majoritaire, La République En Marche, à l'Assemblée nationale. À l'issue de cette première lecture, il ne subsiste que quatre mesures, la principale étant le doublement des peines en cas d'occupation illicite d'un terrain et la création d'une amende forfaitaire délictuelle de 500 euros. La création de cette amende forfaitaire est, certes, une avancée positive que j'approuve, mais celle-ci me semble insuffisante à plusieurs titres. Tout d'abord, l'amende forfaitaire ne s'appliquera que si la commune ou l'EPCI respecte les obligations lui incombant en vertu du schéma départemental. Or, comme vous le savez, les schémas départementaux seront en révision à partir de 2019, ce qui rendra de fait la mesure inopérante dès l'an prochain. Nous ne sommes pas là pour défendre les territoires qui n'ont rien fait, mais, dans de nombreux cas, les collectivités sont déclarées en non-conformité avec le schéma, parce qu'il ne leur manque que deux ou trois places. Pourtant, l'amende forfaitaire ne sera pas applicable dans ces cas. il faut noter que cette amende ne s'appliquera pas aux caravanes. Enfin, élément très important, l'amende ne sera pas répétitive, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, dont la dernière décision date du 30 janvier 2018. Il en résultera que les campements illégaux ne pourront se voir infliger qu'une seule amende, ce qui entraînera un risque fort de sédentarisation et une multiplication des campements illégaux, sans oublier l'insolvabilité très couramment évoquée par ces communautés pour échapper à tout type de sanction financière. Par ailleurs, l'amende forfaitaire ne résoudra pas tous les problèmes, notamment celui des « sauts de puce Aussi, mes chers collègues, face à un problème aussi crucial, nous ne pouvons pas nous contenter de ces maigres avancées. Les élus que nous représentons attendent mieux que cela. Cette deuxième lecture doit être l'occasion d'enrichir ce texte et de tenter d'obtenir des avancées supplémentaires pour doter les élus locaux d'outils efficaces. Nous avons la chance d'avoir entre les mains un texte spécifique, et nous savons tous que cette occasion ne se représentera probablement pas. Nous avons obtenu des garanties très fortes de la part du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale pour que le texte soit inscrit rapidement en deuxième lecture, nous permettant ainsi d'organiser cette navette parlementaire et d'avoir un texte abouti pour la saison prochaine. Aussi ai-je décidé de déposer plusieurs amendements, cosignés par une cinquantaine de mes collègues, visant à rétablir les principales dispositions du texte initial. ces amendements permettra notamment de rétablir un dispositif pour éviter les « sauts de puce », d'autoriser la saisine des véhicules non affectés à l'usage d'habitation pour les transférer vers des aires d'accueil existantes du département, de comptabiliser les aires permanentes d'accueil des gens du voyage sédentaires dans l'évaluation de la proportion de logements sociaux comptabilisés en application de la loi SRU et, enfin, d'instaurer une période transitoire pendant laquelle ces dispositifs pourraient s'appliquer pour une commune ou un EPCI qui aurait cessé d'être en conformité à la suite de la révision de celui-ci. Ces agissements délictueux sont fort heureusement le fait d'une minorité, mais parce que ces agissements peuvent entraver l'activité économique, contraindre l'exploitation agricole, empêcher le bon fonctionnement des services publics, porter une atteinte grave au droit de propriété ou à la liberté de circulation, ils deviennent absolument intolérables pour tous : élus, citoyens, professionnels, agriculteurs, force de l'ordre. Comme le disait l'écrivain et conseiller d'État Eugène Marbeau : « La liberté, c'est le respect des droits de chacun ; l'ordre, c'est le respect des droits de tous. » Plus que le droit, nous avons aujourd'hui le devoir d'agir ! Je vous ai

cette proposition de loi d'une grande partie de sa substance : nous sommes partagés entre l'idée de rétablir le texte tel qu'il était, pour donner une véritable

donne des consignes à ses préfets pour aider tous ces présidents de communautés de communes, en particulier dans les territoires ruraux, à mieux s'organiser,

sont régulièrement confrontées à des campements illicites de gens du voyage. Ils investissent en toute illégalité et dégradent des terrains de foot, des espaces agricoles et, parfois, des sites urbains à proximité immédiate d'habitations, créant ainsi des tensions et des troubles à l'ordre public. La création des aires de grand passage, dont le déficit de fonctionnement est à la charge du contribuable local, n'a pas empêché ces comportements. Bien au contraire, car les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives. Face à cette problématique de plus en plus prégnante, la majorité sénatoriale, à travers le texte de notre collègue Loïc Hervé, a pris une heureuse initiative pour, d'une part, soutenir les communes et leurs groupements dans leur mission d'accueil des gens du voyage et, d'autre part, renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d'installation illégale en réunion sur un terrain public ou privé. Las, comme beaucoup d'entre nous l'ont dit, le texte qui nous est soumis en deuxième lecture est très en retrait par rapport au texte initial. On ne peut que regretter la position de la majorité gouvernementale à l'Assemblée nationale, qui a remis en cause des avancées fondamentales. Je pense, en particulier, aux dispositions qui auraient permis à la fois de faciliter l'évacuation des campements illicites, de renforcer les sanctions en cas d'installation en réunion et sans titre sur un terrain et de condamner les auteurs de dégradations commises à cette occasion. La proposition de nos collègues visant, notamment, à rétablir l'article 5 pour empêcher les « sauts de puce » -évacuations suivies d'occupations d'autres terrains à proximité -aurait toute sa place dans cette réforme, mais, comme le dit le proverbe, « un tiens vaut mieux que deux tu l'auras ». Aussi, je me rallie à la recommandation de voter la proposition de loi dans sa version transmise par l'Assemblée nationale. Nous n'aurons pas pour autant dit notre dernier mot. Nous ferons de nouvelles propositions pour contrer les occupations de terrains non prévus à cet effet. Pour l'heure, il est nécessaire de donner des outils aux maires, qui sont dans une position d'attente très forte.

de supprimer une disposition qui revient subrepticement, clandestinement, à introduire une obligation nouvelle pour les communes de moins de 5 000 habitants, à savoir l'accueil des gens du voyage. du voyage. Si un établissement public où il n'y a que des communes de moins de 5 000 habitants est assujetti à cette obligation, les communes le sont aussi

tout et n'importe quoi. Excusez-moi cette cuistrerie, mais, comme le dit Hannah Arendt, adopter la politique du moindre mal, c'est oublier que le moindre mal, c'est quand même le mal.

les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. La compétence en matière d'accueil des gens du voyage étant transférée au niveau intercommunal, tous les EPCI à fiscalité propre comportant une ou plusieurs communes de plus de 5 000 habitants sont donc soumis

au moment de l'adoption de la loi, la construction d'aires d'accueil dans des communes de moins de 5 000 habitants n'était envisagée que dans le cadre de la coopération intercommunale, et si ces communes de moins de 5 000 habitants étaient comprises dans une agglomération. Il n'a jamais été question d'imposer la construction d'aires d'accueil dans de petites communes rurales. En pratique, il arrive que les schémas départementaux prévoient la réalisation d'accueil en milieu rural, dans des communes de moins de 5 000 habitants, appartenant à des communautés de communes ne comportant aucune commune de plus de 5 000 habitants, mais il est alors précisé dans le schéma que ces dispositions n'ont qu'une valeur indicative

à Mme Sylviane Noël. Cet amendement reprend une disposition du texte initial, qui avait été adoptée en première lecture. Il s'agit de permettre de soutenir les collectivités locales qui s'engagent pour la création d'aires d'accueil en prenant en compte les aires destinées aux gens du voyage sédentaires,

accessibles dans la durée dans des conditions protectrices pour les occupants, qui sont des ménages modestes. La Haute Assemblée l'a d'ailleurs bien considéré ainsi lors des débats tenus récemment à l'occasion de la loi ÉLAN, ÉLAN, rejetant tous les amendements visant à inclure dans le décompte SRU des dispositifs qui ne répondent pas à ces critères pour ne retenir que les logements faisant l'objet d'un bail réel et solidaire et ceux acquis en prêt social location-accession, les PSLA, pendant une durée limitée. Dans ces deux cas de sédentarisation, les conditions d'éligibilité applicables aux ménages bénéficiaires

D'une part, cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour le maire ou le président de l'EPCI de demander au préfet de mettre en demeure les occupants illicites de quitter non pas seulement les lieux mêmes de cette occupation, aussi le territoire de toute la commune, voire de l'EPCI. Ce dispositif est conçu pour lutter contre les « sauts de puce », ces situations où l'évacuation d'un terrain conduit à l'occupation d'un terrain proche. D'autre part, l'article 5 rétabli étendrait les cas où cette mise en demeure peut être prononcée. Jusqu'ici, seuls les troubles à l'ordre public, c'est-à-dire les atteintes à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, étaient concernés. Le vote de cet amendement permettrait d'étendre cette possibilité de mise en demeure aux atteintes significatives au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, afin d'offrir une meilleure protection aux propriétaires et usagers de terrains privés, notamment agricoles. Quel est l'avis de la commission ? Ma chère

Cet amendement, comme vous l'avez rappelé, madame la sénatrice, permettrait en effet au préfet de mettre en demeure les gens du voyage de quitter non pas seulement les lieux, c'est-à-dire le terrain occupé illicitement, mais aussi le territoire de la commune, voire de l'EPCI, sauf les aires permanentes d'accueil, les aires de grand passage et les terrains familiaux situés sur le territoire de la collectivité. Cette disposition est manifestement disproportionnée au regard de la liberté d'aller et venir. Le trouble à l'ordre public justifiant l'évacuation s'apprécie

être acceptée non plus en matière de troubles à l'ordre public. En effet, c'est seulement pour garantir l'ordre public que le préfet peut faire usage de ses pouvoirs de police en la matière. Je vous renvoie d'ailleurs, sur ce sujet, à une décision du Conseil constitutionnel.

Cet article, qui renforce les sanctions pénales en cas d'occupation illicite en réunion d'un terrain, est nécessaire. Les sanctions actuelles n'ont jamais dissuadé les occupants illicites. Si tel était le cas, nous vivrions une autre réalité dans Je regrette cependant que l'Assemblée nationale n'ait pas retenu la saisie des véhicules, qui aurait été l'arme la plus dissuasive pour obtenir le respect du droit.

Dans toutes les matières où elle a été mise en oeuvre, la forfaitisation de la sanction, qui garantit son automaticité mécanique, a assuré son effectivité. Espérons qu'elle produise là le même effet

Noël. Cet amendement vise à rétablir partiellement les dispositions de l'article 6 supprimées par l'Assemblée nationale. Dans le cas d'une occupation illicite en réunion d'un terrain dans une commune en règle avec ses obligations en matière d'installation d'aires d'accueil des gens du voyage, cette mesure permettrait aux forces de l'ordre de transférer le véhicule non affecté à un usage d'habitation vers les aires d'accueil existantes dans le département. Il s'agit là d'une simple éventualité, qui resterait sans doute rare, mais qui

territoire pour y faire enlever un véhicule. En outre, la saisie de véhicules automobiles est déjà prévue par le dernier alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal, à l'exception, vous l'avez précisé vous-même, des véhicules destinés à l'habitation, qui bénéficient de la protection constitutionnelle du domicile. Si tel est l'objectif de la disposition proposée, cette dernière est donc inutile, car elle est satisfaite par le droit existant. L'avis est donc

satisfaite : l'article 2 de la loi Besson prévoit d'ores et déjà un délai de deux ans pour laisser aux communes le temps de se mettre en conformité en cas de révision. Pendant ce délai, elles ne sont pas considérées comme étant dans une situation de non-conformité. De plus, le paragraphe 3 du même article prévoit un délai de prorogation de deux ans sur demande, si la commune a manifesté la volonté de se conformer à ses obligations.

qu'il nous condamne à choisir le moindre, parce que, en choisissant le meilleur, on risque d'avoir, à coup sûr, le pire

dans ce texte, c'est que les gens du voyage ont bien évidemment des obligations. Nous ne pouvons pas accepter qu'ils n'appliquent pas la loi. Pour autant, les collectivités ont, elles aussi, des obligations, et nous devons faire en sorte,

extrêmement vigilants sur le suivi de l'application de la loi. C'est aussi notre rôle constitutionnel ici, au Sénat, de veiller à ce que la loi entre en vigueur sans tarder et produise bien ses effets rapidement- j'ose dire avant la saison prochaine de 2019.

Le scrutin est ouvert.